l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour 2023 j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire sur ce texte ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 24 bis et j'ai un amendement numéro 59 de même la rapporteure, vous avez la parole. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Cet amendement vise à supprimer l'article 24 bis, en effet, celui-ci étant au chirurgien dentiste ou sage-femme aux infirmiers la permanence des soins ambulatoires, la PDSA l'article entend notamment faire en sorte que les infirmiers participe à la régulation si l'idée est intéressante bien sûr et si l'interprofessionnalité doit être encouragé un article additionnel au projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne constitue pas le moyen approprié de délibéré d'une mesure aussi structurante de plus, les modalités de mise en oeuvre du dispositif demeurent largement inconnues à ce stade, les autres professions de santé aura-t-elle vocation à se substituer au médecin de garde, à l'inverse, l'idée de demander à plusieurs professionnels d'assurer simultanément une permanence, quels sont les besoins réels et justifie-t-il une telle présence comment s'assure-t-on de la bonne coordination de ces professionnels et de la qualité des soins et, enfin, et enfin, et nous l'avons évoqué hier soir : quid de la participation et de l'obligation de la participation des médecins généralistes à à la permanence des soins en toute hypothèse, une telle mesure doit faire l'objet d'une concertation en amont les heures d'organisations représentatives devraient être consultés. Madame la présidente, madame la rapporteure, madame la présidente de commission, mesdames et messieurs, bonjour le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement supprimé cet article Madame la rapporteure revient supprimer cet article revient à supprimer l'introduction de la notion de responsabilit collective dans la participation à la permanence des soins tentante, un établissement contenter de ville et qui permet d'apporter la garantie à la population d'un accès aux soins non programmés, elle vise à rappeler que les médecins doivent s'organiser entre eux pour assurer cette permanence est assurée la juste contribution de chacun dans un équilibre entre établissements de santé publics les établissements de santé privés et professionnels libéraux, par ailleurs, vous l'avez évoqué l'élargissement à d'autres professions se fera dans le strict respect des compétences de chacun et sur le déclenchement par la régulation médicale cet été, a par exemple été expérimentés dans le cadre de la boîte à outils, la possibilité d'envoyer un infirmier à domicile du patient sur orienta sus orientation du SAMU, cela peut permettre de réaliser une téléconsultation assisté par exemple et les retours ont été plutôt positifs, donc pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à votre amendement. Merci. Alors, je vais mettre aux voix donc cet amendement qui a de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est donc adopté et l'article est supprimé, amendement 60 madame la rapporteure. Merci madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues. C'est également un article, un amendement de suppression de l'article vingt-quatre 24 alors qu'on ne se méprise pas, ce n'est pas

il nous arrive avec le 49 3 et c'est d'expérimenter l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée introduit par la rapporteure générale à l'Assemblée nationale et dans le même temps, il y a une proposition de loi qui a été déposée mi-octobre à l'Assemblée nationale et qui sera débattu, je crois, vers le 22 novembre et qui parle également d'accès Direct aux infirmières en pratique avancée, j'ai regardé si les termes de la de la proposition de loi étaient les mêmes que l'art se de de l'article 24, il n'en est effectivement c'est pas identique et je trouve dommage qu'à travers le PLFSS alors que c'est un sujet et alors que je suis favorable et je soutiens les infirmières en pratique avancée hé bien on introduit ce ça par voie d'un d'un article qui encore une fois, n'a pas été débattues, c'est de l'organisation des soins ça constitue effectivement cet accès Direct, une mesure structurante qui ne serait pas sans effet sur le rôle de pivot aujourd'hui reconnus au médecin traitant, et plus largement sur l'organisation du parcours des soins si l'accès aux soins constitue un enjeu important, évidemment, il est important de veiller à ce que la répartition des compétences entre professionnels garantissent également la qualité des des soins sur l'ensemble du territoire cette question mérite d'être étudiée de manière transversale à l'occasion justement d'une loi relative à l'organisation du système de soins un article additionnel au PLFSS n'est pas le véhicule approprié et encore une fois qu'on ne se méprise pas sur cet amendement est-ce qu'il ne dit pas surtout. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure, je comprends le l'intérêt de, de, de votre amendement est-ce que vous essayez de de nous dire à travers ça, malgré tout, vous savez que nous avons besoin d'abord d'avancer, de répondre et d'apporter des réponses à nos compris citoyens en en termes d'accès et de au besoin de répondre aux besoins de santé, vous savez que les infirmières de pratique avancée sont en train de se déployer et se déploie de plus en plus donc cet amendement. De c'était l'expérimentation, nous parlons bien d'une expérimentation qui est proposée dans le cadre de cet amendement est réalisé dans le cadre des structures d'exercice elle permettra de pouvoir étudier vraiment les conditions réelles et les impacts éventuels de cette mesure dans le cas précis, elle permettra de prendre en compte les opportunités et les pistes d'amélioration dans les relations entre les IPA et les médecins traitant pour s'assurer d'une organisation du parcours de soins optimale par ailleurs lancer cette expérimentation permettra aussi de dynamiser le déploiement de cette jeune professions dont les compétences cliniques ont été renforcés par une formation universitaire robuste pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à votre amendement. Merci même Guy autant. Oui merci madame la présidente, moi tout en comprenant l'argumentaire de de la rapporteure, je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis plutôt FAP hein, même très favorable en fait à conserver ce cet article voilà c'est un article qui prévoit effectivement une expérimentation, donc d'un accès Direct aux infirmières de pratique avancée, alors on est un dans le cadre de structure coordonnées qui donne quand même un gage de de sécurité et avec un compte rendu de soins transmis par l'IPA au médecin traitant, donc je crois qu'on a quand même qu'à cadrer le cadrer le processus, moi, je voudrais rappeler que les hyper ont fait quand même 3 ans d'études plus 2 ans de spécialisation, donc on est à, on est quand même à 5 ans ce qui leur donne aussi des des compétences particulières, et qu'il est aujourd'hui nécessaire de libérer du temps médical, donc c'est pas inutile de de le redire. Le déploiement de cette profession aujourd'hui, moi je crois que si on fait rien et, rapidement, on va avoir, on a tout un bataillon d'infirmières en pratique avancée libéral qui sont aujourd'hui prêtes à travailler et qui trouvent pas en fait leur place dans la médecine de ville, d'un côté elle trouve pas de place dans la médecine de ville et de l'autre côté les médecins cherchent du temps médical, donc si on on met pas un marqueur fort en leur permettant effectivement de trouver leur place au sein des exercices coordonnés moi je crains que ces infirmières de pratique avancée demain soit de moins en moins nombreux à vouloir se former nous un grand test, on a 783 infirmières en pratique avancée formés sur ces 783 infirmières en pratique avancée, un seul, un seul aujourd'hui exercent à temps plein dans cet exercice d'un de d'infirmiers en pratique avancée, les autres ne trouvant pas leur place dans les exercices coordonné, alors moi je, je crois qu'il enfin je, je pense qu'il faut le maintenir, par contre, si on veut effectivement et être sûr du gage de leur bonne intégration moi je proposais effectivement que les modalités de coopération entre les médecins traitants des exercices coordonnées des maisons de santé et l'infirmière de pratique avancée libéral soit défini déjà le comité de liaison, en fait, il travaille et puis qu'au sein de des projets médical on intègre l'action merci de ces Monsieur Jomier. Merci madame la présidente, je crois qu'on a largement eu l'occasion au cours des dernières années, les uns les autres d'exprimer notre soutien au développement des infirmières de pratique avancée mais tout aussi régulièrement, de pointer le fait que la bonne méthode pour avancer était que les professionnels de santé entre eux négocie l'émergence de nouvelles fonctions pour les uns et pour les autres et que, par ce travail partagé on progresse et on change la situation actuelle qui est une trop grande concentration sur les médecins d'un certain nombre de fonctions, on a vécu des années où la situation a été celle d'un blocage et avec des décisions ministérielles et on se souvient du dernier Plfss, où le ministre de la Santé nous bombarder de dispositions inadaptés. Et là, depuis quelques mois, il se passe quelque chose et moi je salue la mais la nouvelle méthode peut-être je ne sais pas, mais en tout cas les différents ordres se sont mis autour de la table et ont abouti à un texte commun qui ne règle pas tous, mais un texte commun de l'Ordre des infirmiers, des médecins, des kinés, etc pour dire voilà comment voudrait travailler et maintenant c'est l'étape de la négociation conventionnelle, je dis que ce n'est toujours pas l'heure, que le Parlement Vienne adoptée comme ça un dispositif alors que les négociations sont en cours, on en a parlé hier, cette méthode ce PLFSS son grand défaut quand même c'était brouillon d'être brouillon et de donner un sentiment de texte un peu bâclé voilà, non il n'est pas l'heure d'adopter un article sur le rôle des IPA dans six mois les négociations conventionnelles seront terminés, nous verrons ce que tout ça donne : comment les professionnels ont réparti à nouveau entre les tâches et à ce moment-là, si ce n'est pas te 6 pesant, il sera l'heure d'intervenir effectivement. Merci Monsieur Chassang. Madame la présidente, madame Ministre, mes chers collègues, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire, donc Madame Guillotin et puis Bernard Jomier, pourquoi, parce que, à la fois les deux parce que, actuellement, on a besoin de façon urgente dans certains cabinets d'infirmière de pratique avancée et de ça, d'avoir quand même les grandes lignes pour la qu'il y ait une coordination bon la plus la plus harmonieuse possible si vous voulez entre le médecin et l'infirmière de pratique avancée je pense que c'est effectivement ce binôme peut apporter vraiment des choses très bien dans les maisons de santé mais aussi si vous voulez, pour que ce soit complètement terminée, si vous voulez le le le la loi pour que la loi soit vraiment exécutoire, il faut aussi bien sûr consulter les les médecins et les professionnels pour que c'est eux qui décident effectivement ce qu'on doit mettre dans la loi pour qu'il y ait cette coordination mais voit bien, on voit bien comment ça peut fonctionner, ça ne peut fonctionner que s'il y a vraiment une synergie entre le médecin traitant le médecin référent et puis l'infirmière de pratique avancée, c'est quelque chose qui peut être très important pour disons sauver un peu les les maisons médicales où il y a des difficultés. Merci monsieur fit Madame la présidente, madame la Ministre, moi aussi je voudrais soutenir cet amendement de de Véronique Guillotin, pour plusieurs raisons, l'ensemble des débats là depuis plusieurs jours, montre qu'on est dans une situation tout le monde le constate de crise de plus plusieurs sur premièrement, un problème de démographie auquel on essaye de répondre avec la possibilité pour les médecins retraités de prolonger leur activité réorganisation et puis il y a aussi une forme de révolution technologique dans dans la médecine et dans les années qui viendront, il lui faudra revoir les tâches des des médecins, des médecins d'ailleurs qui sont un peu coordonnateur aujourd'hui dans la tâche des médecins, il y a aussi ce dispatching vers vers les différentes vers les différentes spécialités d'ailleurs qu'on impose d'une façon conventionnelle et ce travail là peut être fait par des infirmiers deux ans des IPA pour pouvoir répondre et soulager les médecins c'est dans d'ailleurs dans le même et esprit qu'on a justement imposer le passage chez le médecin généraliste avant d'aller chez les spécialistes et deuxièmement par exemple qu'on essaye d'avoir un un appel pour pouvoir régler les urgences et l'expérimentation des IPA doit permettre de répondre durablement par la suite à cette réorganisation des parcours de santé qui seront bénéfiques pour nos pour les patients et qui seront surtout intéressants pour pour les finances de la Sécurité sociale. Merci monsieur Milon. puisque je suis d'accord avec l'amendement de la commission, mais je voudrais vous alerter sur un problème qui m'a été soumis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les infirmières libérales qui font une formation en IPA trouvent leur première année de formation financée mais pas la deuxième année, donc je souhaiterais que vous puissiez regardez ce sujet j'ai alerté le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais j'aimerais aussi alerter le ministère. Merci Madame Sollogoub Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, je suis très, très ennuyé moi avec cet amendement et sur ce sujet, évidemment, je comprends votre prudence et et on doit toucher l'organisation des soins avec une main extrêmement prudente, malgré tout, il existe des territoires la, la pénurie est telle que la délégation de tâches et vraiment crucial et puis je me mets aussi à la place des des infirmiers et infirmières qui ont ont fait l'effort de faire cette formation d'IPA et qui, à la sortie, on a presque l'impression qu'il a eu un pas en avant et maintenant, un pas en arrière, en tout cas c'est le ressenti, même s'il faut la plus grande prudence dans l'organisation, moi, moi je, je, je rejoins la la position à titre personnel de de Madame Guillotin. Merci monsieur Cabanel. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, moi je ne suis pas un spécialiste de la santé, et depuis le début de de ces débats, je, je, je, je, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se passe et monsieur le ministre, hier, nous a expliqué qu'effectivement des décisions avaient été prises par le passé qui nous amène dans cette situation aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons et je pense que pour ne pas renouveler les erreurs du passé, je suis dans tous les domaines d'ailleurs pour l'expérimentation et c'est pour ça que je soutiendrai l'amendement de ma collègue Véronique Guillotin, parce que je pense que c'est par l'expérimentation que l'on pourra décider ce que pourra, on pourra mettre Merci madame la présidente de Roche et après, madame la ministre. Oui, moi je voulais dire que pourquoi la commission a pris cette position, bien évidemment qu'on soutient les hyper, je veux dire quand on a fait le rapport sur la commission d'enquête d'hôpital on on a bien mis dans nos propositions, qu'il fallait arriver à ce partage quand la ville va mal, l'hôpital va mal et si on veut en effet que la ville allait bien et deux dé facto soulage l'hôpital d'entrée ou de consultations dans les services hospitaliers, c'est pas ce qu'il faut qu'on est en effet un accès aux soins qui soit le meilleur possible, ça aurait territoire on a eu le débat hier, nous ce que nous voyons dans cette, dans cet article, c'est certes une expérimentation qui fait qu'il est recevable otite du PLFSS mais néanmoins, on est sur une organisation des soins les hordes se sont entendus pour essayer de trouver des propositions mais quand les autres se sont entendus, ce ne sont pas que les IPA donc où entrait dans le PLFSS de tout ce qui peut être en effet des expérimentations pour répondre à ce que dit le Clio et on met tout, mais pourquoi ne le focaliser que sur une profession, alors que c'est quelque chose qui regroupe l'ensemble des professions médicales et paramédicales et et qu'on nous dise pas que qu'on protège les médecins en faisant ça, ce n'est pas vrai, moi j'ai toujours milité pour qu'il y a en effet un partage et qui est un parcours du soin avec le médecin, tous les professionnels de santé autour et c'est beaucoup plus large que les seuls les seuls infirmiers, même s'ils ont une place considérable et et remarquable dans le dispositif, mais cet cet amendement enfin cet article se focalise uniquement sur une expérimentation sur les CPA alors que le problème est beaucoup plus large et pourquoi on a dit qu'on ne le Ross sortait parce qu'il y a, alors on verra si ça passe, mais il y a pour l'instant sur le site de l'Assemblée nationale, inscrit à l'heure du jour une PPL

pour avoir le meilleur accès aux soins la meilleure prise en charge d'un patient sur un territoire ce pourquoi nous renvoyons à un texte en effet si la PPL n'étaient pas étaient sortis de l'Ordre du jour à l'Assemblée nationale, moi, je crois, on travaillera pour qu'il y a quelque chose qui soit fait parce qu'on ne peut pas mélanger, organisation des soins des des articles de PLFSS comme ça disparates, à chaque fois, l'an dernier, on a eu, on a eu les kinés, on a des orthoptistes, maintenant on a les IPA hé hé, et c'est pas du tout contre les infirmiers je le président de l'ordre à, à cet égard, bien évidemment qu'on soutient, chacun a sa place, tout le monde voit bien comment travaillent les infirmiers comment les médecins travaillent sur un territoire avec leur infirmiers avec leur pharmacien avec leur qui naît avec, avec toutes ses promesses avec les sages-femmes et toutes ces professions, donc voilà la position de la commission, en rien dire on balaye d'un revers de main, cette solution, c'est pas non plus pour ça traîne des années, je pense qu'il faut très rapidement cette organisation des soins, elle se fasse entre les différents professionnels de santé mais je valide la position de la commission et je la confirme. Merci madame la Ministre. Moi, je valide la le l'avis défavorable du gouvernement sur vraiment, je le redis je crois et j'en suis intimement convaincu personne ici ne dit que nous n'avons pas besoin des IPA merci madame la présidente, madame la rapporteure de l'avoir redit simplement, nous sommes dans une situation où. Cet article il prévoit quoi, il prévoit une expérimentation cette expérimentation, elle a d'abord la volonté d'être effective, assez rapidement, nous parlerons sur l'amendement suivant des enjeux du client, je vous en parlerai juste après mais cette expérimentation, elle pourra être mise, j'allais dire en oeuvre assez rapidement et cette expérimentation, elle a aussi la volonté de dire que nous avons besoin et nous avons encore besoin, monsieur le sénateur millons d'accélérer sur la formation des IPA donc accélérer sur la formation des IPA c'est d'abord leur faire confiance, l'enfer par confiance dans le binôme médecin IPA, le président de l'Ordre des médecins que j'ai vu hier nous a encore demandé, il nous a encore inciter à aller encore plus vite sur la formation des IPA, donc il faut le déconnecter et j'entends le côté superposition des dispositifs mais c'est aussi un signal très fort que nous envoyons à ces infirmières de pratique qu'dont nous allons avoir besoin très fortement et c'est aussi l'idée de les inviter et d'un d'inciter très fortement les infirmières en ayant un sujet sur les enjeux de prise en compte de la formation et il est réel, mais assez inéquitable entre toutes les régions, donc on a aussi un sujet sur la prise en compte des régions, de pouvoir les les inciter fortement à se former, je crois que c'est un signal fort et nous devons aussi envoyer des signaux forts à certaines professions, nous avons besoin des infirmières, nous avons besoin des infirmières de pratique avancée et nous devons lancer cette expérimentation qui viendra compléter le dispositif sur lequel nous sommes encore d'en train de travailler avec le Clio mais je vous en dirai un mot sur l'article suivant, donc je pense que nous devons avancer, c'est pour ça que le gouvernement maintient son avis défavorable sur l'amendement de Madame la rapporteure. Ah si Monsieur Savary. Oui, vous voyez, Madame la Ministre, moi j'ai, j'étais un peu dans le doute, mais maintenant, vous m'avez convaincu que de soutenir l'amendement de Madame le rapporteur, ben oui, vous voulez donner des signaux, des images de la communication, très bien, c'est bien les difficultés qu'on peut rencontrer, nous on veut une vision et la vision à, doit être pris par les partenaires sociaux, par exemple en ce qui concerne la branche vieillesse et les retraites, elles doivent pris par les ordres et les syndicats médicaux en ce qui concerne l'organisation des soins c'est un PLFSS on va pas refaire tout l'organisation des soins à travers ce PLFSS ou alors madame la ministre est chez vous, a présenté une loi santé d'organisation, qu'ils soient là véritablement la réponse partagé par l'ensemble des professionnels et des usagers pour répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer, donc moi j'ai envie de mes collègues à soutenir cette proposition qui est là juste proposition, il doit y avoir des conventions, hé ben c'est à ce niveau-là, mais par contre, s'il y a pas de résultats dans les conventions, sachez qu'on saura prendre nos responsabilités. Merci monsieur lévrier. et à partir du moment où on parle pas d'une expérimentation, je m'étonne de des réactions sur certains bancs à ce sujet-là, parce que je pense qu'un sujet très important et qu'on doit effectivement montre des signaux, même et surtout à travers le PLFSS. Merci, alors je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

alors 3 E trois amendements faisant l'objet de d'une discussion commune et je vous dis que l'amendement 1020, a été retiré avant la séance, alors là, mon nom 61 madame la rapporteure. Merci madame le président, madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement concerne l'organisation des consultations avancées, sujet qui a été abordé hier soir une telle expérimentation procède des recommandations du rapport charges produit de la CNAM, que son directeur général nous avait présenté en en commission en en juillet dernier, cela contribuera utilement avec la rationalisation des aides à l'installation engagée par l'article 24 à remédier aux conséquences de la faible démographie médicale donc cet amendement réécrit, hein, un tout petit peu, l'article 24 quater mais sur le fond, ce voilà ça me favorable. Merci madame la Ministre pour le sous-amendement. Donc le gouvernement donnera un avis favorable à la maman de de Madame, la rapporteure, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qui souhaitent garantir l'uniformité de la rémunération des consultations avancées entre les régions. Merci l'amendement 1096 Monsieur Jomier. Merci madame la présidente, donc effectivement on a eu, on a commencé le débat hier, donc je je vais être bref, oui, il faut mettre en place ce type de dispositif la rédaction initiale le confier intégralement aux heures des médecins, ça n'était pas une bonne chose, la rapporteure, a présenté une position qui inclut maintenant les ARS, enfin qui élargit le le type d'organisation, c'était ce que prévoyait notre amendement est donc je le retire. Monsieur bonne. Hein madame Jacques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est un amendement de notre collègue Florence Lassaad cet article prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de 3 ans de l'État peut autoriser le Conseil de l'Ordre des médecins, territorialement compétent organisé obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones déficitaire en offre de soins dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ses médecins la coercition ne permettra pas de régler le problème de l'accès aux soins, en revanche, l'incitation doit être la règle pour valoriser ses consultations avancées là où elles sont nécessaires. Merci l'avis de la commission, même le rapporteur. Merci, M. le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un avis favorable de la commission sous-amendement du gouvernement donc l'amendement, monsieur, je m'y été retiré et c'est une demande de retrait, à défaut d'un avis défavorable pour l'amendement 300 337. Merci l'avis du gouvernement. Qu'une demande de retrait pour les 2 amendements 1096 et 337 profite du l'amendement 61 pour lequel l'amendement sous-amendé par le gouvernement, nous avons donné un avis favorable.

je vais passer la parole à Madame Guigou, autant pour le 583. Merci madame la présidente, je peux te présenter les deux en fait fait office d'amendements et quelque part de sous-amendements, voilà, moi je suis père favorable et très contente que le le l'amendement l'article précédent soit a été été adoptées donc pour l'expérimentation effectivement de certains médecins qui puisse aller exercer en zone plus difficile ou en zone sous-dense alors effectivement là d'hier, à un moment donné, c'était interdit, aujourd'hui on est obligé de revenir sur la loi, mais bon, les conditions sont sont ainsi et je crois qu'offrir cette liberté-là, au médecin est une bonne chose, mon amendement demande pour aller encore plus vite et plus rapidement que cette expérimentation soit donc dans le 583 sur l'ensemble du territoire national et en amendement de repli 594 pour étendre à 6 régions au lieu de 3 l'expérimentation précédente. Merci le 889 monsieur lévrier. Merci madame la présidente, et je souhaiterais par cet amendement va nous c'est par cet amendement que l'expérimentation s'étendent à au moins un territoire ultramarin, qui est ce qui nous paraît aussi très important merci beaucoup. Merci l'avis de la commission, même la rapporteure. Merci madame le président, madame la ministre, chers collègues, alors cette année à une demande de retrait des fois un avis défavorable sur le 583 c'est un avis favorable sur le 594 qui étend l'expérimentation à 6 régions et c'est un avis favorable sur le 800 89 qui souhaiterait qu'un territoire ultramarin au moins soient concernées par cette expérimentation. Le gouvernement s'remet à la sagesse des sénateurs. d'accord merci donc je mets aux voix le 594 qui a reçu un avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement qui, pour qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté le 800 89 a même avis même vote

Merci madame la présidente, à la mise à disposition de personnel par des entreprises de travail temporaire, ces dernières sont d'ailleurs mais à tort considérée comme l'une des causes des pénuries de personnel alors qu'elle ne représente qu'une part minoritaire de mise à disposition de personnels de santé dans les établissements de santé et qu'elle contribue à la continuité des soins, en particulier dans les déserts médicaux, d'autres formes de mise à disposition de personnels qui sont certes moins connue, mais qui existent et qui sont proposés par d'autres, ce type de structures comme les sociétés coopératives des groupements d'employeurs, les entreprises travaillent à temps partagé, doivent également être concernés par cette régulation et non le seul travail temporaire au sens strict, le gouvernement a également précisé que les dispositions envisagées concernés, les jeunes diplômés particulièrement sensible aux conditions de tutorat lors de leur première prise de poste et à la sécurisation de leur transition professionnelle et qu'il s'agissait de renforcer la régulation de l'intérim, en début de parcours professionnel, c'est pourquoi le présent amendement précise que les personnels de santé concernées par l'article 25 sont ceux qui n'ont jamais été mise à disposition auprès d'un établissement de santé, à défaut, cela signifierait que les dispositions prévues par l'article 25 s'applique à tous, personnel de santé, qu'il soit en début de carrière ou non, donc ce serait à leurs contraires à l'objectif affiché par le gouvernement dans l'exposé des motifs de l'article 25 ainsi qu'à l'étude d'impact de cet article dans le PLFSS qui indiquait que cette mesure favorise favorisera donc l'orientation des jeunes professionnels vers un premier emploi en établissement de santé afin qu'ils y acquièrent une solide expérience. Merci madame la présidente, l'amendement que nous présentons, vise à renforcer le dispositif proposé en étendant la condition de durée minimum d'exercice dans un cadre autre que des missions d'intérimaires aux professionnels de santé, mise à disposition auprès d'un établissement de santé situés en France ayant un contrat conclu par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger sans cette mesure, il y aurait un manquement pour ce cas très précis de de professionnels de santé ayant un contrat avec une entreprise à l'étranger, cette situation existe et nous le savons, il faut donc répondre à celle-ci et s'assurer que le dispositif intègre ces contrats, c'est l'objet de cet amendement, merci. Merci, il le 1015 filleule oui madame là. Présidente, Madame la Ministre, cet amendement vise à étendre la régulation imposée aux intérimaires, aux soignants, passant des contrats de gré à gré en effet réguler l'intérim 100 réguler les contrats de gré à gré, rendrait l'article 25 inefficace, le recours à l'intérim médical pèse lourdement sur les finances des établissements de santé, annuel a explosé pour l'hôpital public, passant de 500 millions d'euros en 2013 à un milliard 4 d'euros en 2018, une étude de la Direction générale des finances publiques d'octobre 2021, nous indique que le taux de recours au travail temporaire pour le personnel médical atteint près de 20 pour 100 ce chiffre important incluent l'intérim médical strict et les contrats de gré à gré, cette pratique est dénoncée de longue date, notamment par la Fédération hospitalière des hôpitaux publics si nous légiférons seulement sur les contrats passés par le biais des entreprises d'intérim alors les intérimaires se reporteront vers les contrats conclus de gré à gré, c'est pourquoi le présent amendement vise à garder l'esprit de cet article en protégeant les hôpitaux de la surcharge financière que représentent les intérims dans l'hôpital public, merci.

je comprends bien sûr les les arguments de notre collègue Dominique Estrosi Sassone. Sur le fond, limiter l'interdiction aux entreprises de travail temporaire pourrait paraître insuffisant cependant le champs des entreprises de travail à temps partagé ou des plateformes que l'amendement visés sont mal identifiés par ailleurs dans les groupements d'employeurs qui serait exclu, je m'interroge sur les risques possibles que pourrait produire une telle exclusion des groupements d'hôpitaux ne pourraient ainsi se constituer pour s'organiser collectivement et ça c'est quand même relativement dommage pour ces raisons, et devant les incertitudes qui sont non négligeables, hein, dans ce domaine, il a semblé à la commission qu'à ce stade d'évolution du Champ d'interdiction n'était pas opportun, j'aurais cependant une question à vous adresser, Madame la Ministre, nous entendons tous lutter contre l'intérim médical, pouvez-vous nous éclairer sur le nombre de contrats d'intérim, le nombre de mises à disposition relevant d'autres types d'entreprises que des entreprises de travail temporaire parce que c'est bien là le sujet, comment se répartissent les volumes et les parts de marché du secteur et enfin concernant les sociétés organisant de telles mises à disposition combien celui qu'Élysée en France, où sont situés les entreprises de ce secteur établis à l'étranger, ce qui est un vrai sujet également là dessus, voilà sur un dernier point juste la rédaction de l'amendement prévoit d'exclure du Champ et donc de permettre l'intérim aux professionnels en ayant déjà fait et d'ayant déjà fait de telles missions d'intérim, si je prends un exemple : un infirmier avec 2 ans de pratique sans intérim. Pourrait être interdit quand un un infirmier avec quelques mois de pratique seulement mais il déjà fait de l'intérim serait encore autorisés en faire, voilà donc il y a un petit problème de de rédaction, donc c'est plutôt demande de retrait des fois on a un avis défavorable en l'état. Sur l'ensemble, même ma mère important. Alors l'amendement 894 je reconnais à notre collègue Martin lévrier un souci certain de la qualité de de la rédaction de de la loi et je l'en remercie donc ces précisions rédactionnelles sont bienvenues, c'est un avis favorable, madame. Et sur l'amendement 1015. la question est pertinente, je me suis interrogé sur l'opportunité de l'extension du Champ d'interdiction, contrat de gré à gré, j'ai posé cette même question fédération hospitalière, cela ne leur sont pas opportun pour des raisons assez clair qui m'ont conduit à ne pas proposer cette extension et qui ont conduit la Commission a donné un avis défavorable, d'une part ce que l'on appelle le gré à gré, et mal défini s'agit en réalité du droit commun, encadrés par ailleurs ces contrats ont des plafonds définis et inférieur aux contrats d'intérim, d'autre part et surtout, il faut bien voir que ces contrats sur la forme qui permet de rentrer dans les hôpitaux, si je peux me permettre expression c'est par le biais de contrats Directs avec les établissements que se prépare le concours de praticien hospitalier, par exemple, et c'est par le biais de tels contrats que sera aussi demain rempli la condition que l'article 25 imposent pour accéder à l'intérim, donc à défaut d'un retrait, c'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Si vous me permettez, la présidente, je vais répondre et donner quelques chiffres concernant l'intérim tout d'abord pour dire que. Pour l'hôpital public, le coût annuel de l'intérim est passé de 500 millions d'euros en 2013 à 1424 millions en 2018, nous ne devons pas encore les chiffres consolidés là mais ça ne fait encore qu'augmenter ces dernières années pour les personnels médicaux, les dépenses d'intérim donc des personnels intérimaires, via une entreprise de travail temporaire sont passés, eux, de 167 millions en 2021 contre 162 millions en 2019, ces données sont des données comptables extrait des Budgets des établissements publics de santé, on voit bien que le recours à l'intérim dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux n'a cessé de croître au cours des 2 dernières décennies, le recours à l'intérim, a plus que doublé de 2000 à 2021 dans les établissements de santé, et a été multiplié par 10 dans les établissements du secteur social et médico-social, et médico-social, ce qui nous inviter, nous inciter à réagir. Attention. Madame Estrosi Sassone pour votre amendement le Gouvernement émet un avis défavorable, votre amendement propose d'élargir le dispositif, donc de l'article 25 à toutes les formes de mise à disposition de personnels autre que celles réalisées via une autre ville de travail temporaire, nous partageons tous l'objectif de régulation des dérives de l'intérim médical mais votre amendement ainsi rédigé appelle plusieurs observations tout d'abord la notion de mise à disposition de personnels mérite une caractérisation précise à fortiori si elle est inscrite dans la loi, en effet, cette notion recouvre notamment une position statutaire pour les agents publics titulaires de la fonction publique et pour les patriciens hospitaliers vous évoquez par ailleurs des sociétés coopératives groupement d'employeurs et entreprises de travail à temps partagé, sans préciser clairement le statut des entreprises que vous souhaitez visé et soumettre aux dispositions du présent article 25 il en résulte un flou sur l'objet de l'amendement et l'objectif poursuivi pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement. Pour l'amendement. 894 pour les mêmes raisons que le rapporteur, un avis favorable. Et pour l'amendement mille cinq de même Madame filleul pour les mêmes raisons que la rapporteur un avis défavorable, le gré à gré en porterai plus de problèmes que de réponses. Merci, alors j'ai 2 mondes pour Monsieur Chassang. La présidente, madame la miss, mes chers collègues, bon ça va pour moi très rapide, je voulais quand même indiqué qu'il faut régulariser d'intérim mais dans les EPHAD alors c'est pas dans les déserts médicaux, c'est dans des endroits où il y a des Epad qui sont un peu loin, parfois un peu loin des des villes moyennes ou des ou des CHU s'il n'y a pas d'infirmières intérimaires, on ne fonctionne pas, merci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix, alors le 390 a été retiré, madame Estrosi Sassone merci le 894 avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient et donc adopté et le 1015, qui a reçu un avis défavorable de la commission défavorable du gouvernement qui est. Pour qui et contre qui s'abstient une maison pas adopté l'amendement 907 Me Poncet mon Merci madame présidente alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux sociaux contribue pour une large part à leur formation, une grande majorité de ma soeur, qui n'hésitera peu d'orthophonistes, d'ergothérapeutes et de motricien souriant dès leur diplôme obtenu vers un exil exercice libéral, or cette situation, ajoutée à celle d'un numerus clausus faible mais en grande difficulté, de nombreux établissements les postes non pourvus au sein des établissements contribue à étendre les zones sous-denses en spécialiste dans certains territoires ainsi selon l'adresse en 2019, 75 % des habitants en territoires ruraux ont des difficultés d'accès des ma soeur qui n'hésitent thérapeute concomitante à la pénurie de généralistes, la pénurie de spécialistes de paramédicaux constitue un problème majeur d'accès inégal aux soins et freine l'installation d'autres professionnels de santé dans un cercle qui est devenu vicieux cet amendement propose donc de conditionner l'installation en libéral des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens une durée minimum d'expérience professionnelle au sein d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service social ou médico-social. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. avant que nous envisagions un un élargissement voilà demande de retraite. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Une demande de retrait sinon un avis défavorable pour les mêmes raisons que la rapporteure. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 900 cet avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour,

de santé cependant, alors que l'intérêt médical et paramédical fragilise dangereusement les équipes de soins, la préservation de la qualité de centre de soins passe pour tous et pour tous les professionnels, au-delà des seuls jeunes diplômés par une pratique en activité stable le présent amendement vise ainsi à ce que l'intérim ne soit ouvert dans le cas de contrat de mise à disposition, qu'à des professionnels ayant exercé récemment dans le cas de contrat classique même à durée déterminée, l'article entend permettre une exigence différentes selon l'ancienneté des professionnels dans leur exercice et préserver l'intention d'interdiction aux jeunes diplômés à cette fin, d'appréciation de la durée d'exercice sur les 12 derniers mois, tient compte de l'exercice préalables. Merci le 325 qui le défend même Jacques. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, le recours à l'intérim représente pour les établissements hospitaliers, un coût non négligeable qui grève considérablement leur budget, outre son impact financier majeur dans les Budgets des établissements de santé, le recours à l'intérim médical engendre également une déstabilisation des services hospitaliers, les équipes médicales et soignantes susceptibles de nuire à la qualité des soins, de surcroît, le recours à l'intérim est un facteur de tension, les praticiens qui s'investissent durablement dans le service public hospitalier se sentent dévalorisés vis-à-vis de médecins de passage aux rémunérations sans commune mesure avec les leurs, cet amendement vise donc à réguler un peu plus le recours à l'intérim, en limitant à une durée de 5 ans, la période d'intérim dans une carrière.

ça l'amendement qui ne pas contre l'intérim effectivement médicale mais qui vise à éviter un certain nombre d'abus ou d'aspects négatifs à fonctionnement à travers cet intérim qui s'est vraiment développée et a pris des proportions qui aujourd'hui génère des coûts qui sont injustifiées fragilise les finances de l'eau établissements conduisent à ce qu'il y a une insuffisance ou voire un manque d'implication dans les établissements et en tout cas une moindre participation aux équipes soignantes dont on sait que c'est une des conditions de la qualité des siens, des soins, pardon, ça génère également une équité entre des personnels qui exercent des, des, des mêmes missions au sein d'un d'un établissement, puis d'une certaine manière, on le constate un effet boule de neige, puisque des personnels par je passe d'activité sous statut à des activités intérimaire, néanmoins, nous avons besoin de de cet intérim d'abord pour répondre à des sur le personnel de professionnels de santé qui peuvent avoir besoin temporairement d'être dans ces situations d'activité et puis également pour répondre aux besoins de nos établissements, mais il s'agit d'en d'en ah d'assumer une une activité d'une régulation de cette activité là et c'est la raison pour laquelle les proposer de limiter à 6 mois sur des durées et des périodes glissantes de 5 ans cette possibilité d'exercer des intérims, cette période de 6 mois est porté à 24 mois pour les établissements situés dans des zones sous-dotées, je vous remercie. Mais si l'avis de la commission madame la rapporteure. Sur les amendements 325 et et 421 ce serait une demande de retrait au profit de l'amendement de la la commission, il est clair qu'on ne fait pas carrière en en intérim, je pense que la rédaction des amendements me semblent ne me sens pas opérationnels et voilà c'est pour ça que je vous propose de retirer votre votre amendement, mes chers collègues, au profit de l'amendement de la commission. Merci l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements donc chacun avec des axes différents, nous sommes tous d'accord qu'il faut lutter contre l'intérim, l'objectif de cet amendement, hé bien de donner une durée globale unique apprécié dès le début de la carrière qui paraît plus adapté l'amendement notamment déposé par la commission, l'amendement 62. Limiter l'appréciation de la durée d'exercice maximale 12 derniers mois restreint excessivement le Champ d'application du présent article et surtout complexifie

Merci madame la ministre, hein, alors je vais mettre aux voix l'amendement 62 qui étonne même Jacques il est retiré, merci, donc l'amendement 62 de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est. Pour qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté l'amendement donc 421 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, contraint qui s'abstient donc pas adopté l'amendement 63 madame la rapporteure. Merci madame le président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'extension de l'interdiction du chant des établissements sociaux et médico-sociaux a été assortie d'une possibilité de de sanctions, en vue de garantir le respect de de cet article, il convient de prévoir également des sanctions au sein des dispositions propres aux établissements de santé, telle est l'objet de cet amendement.

or le présent article de loi prévoit déjà que ses modalités d'application sont fixées par décret cette mention recouvre notamment les sanctions applicables en cas de non respect de l'interdiction posée par la loi, dont les modalités doivent être encore définis, l'amendement étant déjà satisfait propose un retrait sinon avis défavorable. rapporteure. Oui, madame la présidente, madame le Ministre oui comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, il faut essayer de limiter l'intérim mais attention aux sanctions parce que

merci madame le président, j'ai bien entendu l'avis défavorable de Madame la Ministre, mais nous ne faisons qu'harmoniser la rédaction, rien de plus là loin en prévoyant des sanctions concernant l'intérim dans le Champ des établissements de santé, ni plus ni moins. La rédaction a été voilà hein, c'est la rédaction du gouvernement, nous ne faisons harmoniser ce qui est écrit. Merci, alors je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu, donc un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contraint qui s'abstient, il est donc adopté l'amendement 64 madame la rapporteure. Merci madame le président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rôle de l'Agence Régionale de Santé doit être renforcée en appui aux établissements de santé, en vue d'apporter une réponse coordonnée et cohérente à l'échelle du territoire, la commission souhaite que les ARS puisse assurer une mission de soutien aux établissements permettant à ceux-ci de lui déclarer des besoins en personnel de nature à remettre en cause leur activité la res aurait pour mission d'appui les établissements priorisant des demandes au regard des besoins sur le territoire, elle pour en amont s'assurer d'un vivier de renforts disponible en lien avec des sociétés d'intérim aussi de la mission de soutien à la continuité et à la qualité des soins du fonds d'intervention régional financer certains contrats, les contrats demeurerait conclu à l'initiative des établissements, l'ARS n'ayant pas vocation à se substituer. Merci l'avis du gouvernement, Madame la ministre. le gouvernement émet un avis très défavorable sur cet amendement, tout d'abord la première partie de votre amendement existe déjà dans les faits, les ARS connaissent de manière fine les difficultés des établissements et adaptent leur réponse en fonction de ses difficultés, l'article L 14 31 2 prévoit déjà ce rôle dans l'observation de la situation de la région et la situation et la gestion des situations de crise, la seconde partie prévoit la mobilisation du firent un outil souple, géré par les ARS qui oriente les financements vers les besoins identifiés des territoires un fléchage tels que celui envisagé n'est pas nécessaire par ailleurs votre amendement ne correspond pas à l'objectif de la politique que nous menons en la matière qui est d'encadrer l'exercice professionnel en intérim et de stabiliser les collectifs de travail pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable. Merci madame la présidente, je je profite pour expliquer notre vote au niveau donc de notre groupe, parce que, effectivement, je crois qu'on est tous d'accord, par rapport aux effets négatifs de l'intérim après on essaye, me semble-t-il, de bricoler un certain nombre de, de, de mesures qui ne sont pas vraiment toutes satisfaisantes, il faudrait reprendre les choses de manière plus globale, je voudrais vous dire madame la ministre, et vous le savez que Monsieur Brom, d'ailleurs, a dénoncé lui-même l'intérim cannibales et il a dit que ça risquait de fissurer profondément l'esprit d'équipe chez soignants et c'est vrai que, en même temps, alors que, il y a un manque criant de de soignant l'hôpital certains médecins effectuent des missions temporaires qui font monter les enchères jusqu'à quatre mille euros la garde et, selon la Fédération hospitalière de France, l'intérim médical représente 10 milliards d'euros pour les les hôpitaux il y a un décret effectivement de 2017 qui encadrent le travail intérimaire dans les hôpitaux, à 1100 5170 euros la garde de 24 heures pour un médecin, mais j'aimerais vous demander, Madame la Ministre,

l'on l'on pose avec ma collègue, Céline Brulin, et c'est extrêmement important parce que, comme ça n'est pas respectée, hé bien il y a une mise en concurrence entre les établissements, parce qu'il y a un manque cruel de de personnel et ça fait monter encore les les enchères, je citerai Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, selon lequel il faut immédiatement réguler ce travail intérimaire avec l'accès avec l'arrêt pardon de ces salaires mirobolants et dans le même temps revaloriser les gardes hospitalières et vu le temps qui m'a un parti j'attire votre attention madame la Ministre, si vous m'écoutez sur cette revalorisation, qui n'a pas été fait depuis 20 ans, 250 euros c'est vingt euros de l'heure pour quelqu'un qui a fait 10 ans d'études. Donc, mais il faut aller merci, cher collègue, alors je mets aux voix donc l'amendement 64 de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté je mets aux voix, l'article 25 et pour qui compte qui s'abstient et donc adopté après l'article 25 1062 Madame Jasmin. Merci madame la présidente, madame la ministre, cet amendement concerne les outre-mer et particulièrement les problématiques liées au coefficient tu es géographique, la Fédération hospitalière de la Guadeloupe, présidé par le Docteur André Atallah, qui est cardiologue m'encore alerté il y a quelques jours, alors la crise sanitaire, a mis en lumière les difficultés structurelles de l'offre de soins en outre-mer et les sous-dotation généralisée dans les établissements concernés depuis plusieurs années, nous alertons le gouvernement sur l'urgence de revoir le financement de cet établissement et notamment par la revalorisation du coefficient géographique car dans tous les établissements des outre-mer il y a vraiment des surcoûts qui sont liés à l'insularité à l'accréditation à la certification à l'amélioration continue de la qualité et aussi et surtout aux difficultés liées aux stocks tampons parce que vous n'avez pas les mêmes problématiques sur le territoire hexagonal, alors que chez nous, il faut le haut des steaks, des stocks tampons et avec la situation sanitaire, il y a eu de grosses pertes également parce que tous les examens n'étaient pas faits par exemple les laboratoires et les les services supports doivent aussi avoir la qualification des équipements, ce qui est nécessaire, alors qu'ici il y a des coûts s'est amplifié sur nos territoires les évacuations sanitaires également parce que nous sommes par exemple en Guadeloupe, un archipel mais l'ARS de Guadeloupe, c'est aussi, c'est Martin et ses Barthélemy, et la plupart du temps il y a beaucoup d'évacuation sanitaire, ce qui augmente les surcoûts, donc je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous puissiez prendre en compte les difficultés de ces territoires, à cela s'ajoute tout ce qui concerne la mise aux normes des de certains établissements par rapport aux risques naturels majeurs et aussi les difficultés liées au impersonnel, parce que là vous avez, vous venez de parler des personnes qui viennent travailler en intérim, mais chez nous on les a pas vraiment, ce sont des personnes, en fait, bon je vais pas dire parce que c'est des surcoûts considérables, des personnes qui travaillent ici, qui viennent travailler là-bas ça rend service, c'est vrai, mais pour quel prix les établissements sont confrontés à c'est sûr qu'on l'a également, et les prix, je voulais savez mieux que moi, l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci madame le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article du code de la sécurité sociale que cet amendement modifie prévoit déjà que des coefficients géographiques s'applique et, je cite, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste permanentes et substantielles, le prix de revient de certaines prestations, la situation des outre-mer et bien évidemment préoccupante mais la rédaction actuelle ne se trouverait pas amélioré par les précisions de cet amendement qui, une demande de retrait des fois un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. madame la présidente, madame la sénatrice bien sûr l'outre-mer nous occupe et nous préoccupe, je suis d'ailleurs aller à la Réunion et ce sujet sur le coefficient géographique a été évoqué par vos collègues là-bas je vous rappelle néanmoins que le le. Coefficient géographique vise à compenser certains spécifiques qui sont liés à la zone géographique, et plus particulièrement à l'insularité à l'éloignement parmi les postes de surcoût identifié est liée à la zone géographique que le surcoût du personnel que vous avez évoqué le prix d'achat des médicaments auxquels s'ajoutent les frais d'approches et d'acheminement par exemple, soucieux de prendre en compte la réalité des surcoûts sur supporter sur ces territoires, le gouvernement a confié l'an passé à la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, l'adresse une étude relative au calcul des coefficients graphique, ces travaux sont encore en cours et doivent ta bouche aboutir prochainement, il me semble utile à ce stade, de ne pas modifier les termes de la loi, en attendant les résultats de ces travaux, donc, pour cela, nous demandons une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 1062 monsieur je oubliais pardon. Oui merci, quelques mots, madame la présidente, parce que depuis des années, ces questions sont soulevées et depuis des années, ce sont les mêmes réponses des ministres qui oui c'est pas vous faire un un jour, je Madame la Ministre, ce ce, ça ne vous concerne pas personnellement, mais à chaque fois les ministres nous font exactement le même type de réponse, moi je veux juste attirer l'attention sur un point, c'est que toutes ces questions soulevées sont des questions juste voyez, nous n'y répondons pas depuis des années et que le résultat c'est que lors des derniers cycles électoraux, ce sont les parties les plus protestataires qui ont recueilli les votes des électeurs de ces départements, tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'abandon qui ne nourrit que de la colère et du rejet de ceux qui gouvernent le pays, voilà donc l'amendement de Madame Jasmin, si on l'adopte ne réglera pas le problème, on en est bien d'accord, mais c'est plus qu'un amendement d'appel, c'est un amendement d'appel au secours. John anniversaire. Franchement, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est bien parce que l'étude de l'adresse a été lancé et que, une fois le rapport de cette étude c'est assez compliqué, hein, je peux vous assurer pour un maître penché lorsque je suis allée à la réunion sur l'enjeu de ces coefficients géographiques, avec tout ce qui les impacts, c'est bien parce que cette étude est lancée, qu'elle est complexe qu'il faut le lui laisser le temps d'être faite et une fois que le que les résultats seront connus, nous prenons l'engagement bien sûr de travailler avec tous les acteurs du territoire, une fois les études de les résultats de cette étude connue, l'étude est lancée, nous ne faisons pas rien la problématique elle est réelle et c'est bien parce que la problématique elle est réelle, qu'il nous faut attendre les résultats de cette étude et que nous pourrons travailler sur la base des résultats produits. Merci monsieur Milon. merci madame la présidente, je je voterai l'amendement pour une raison simple, c'est que nous avons fait une mission il y a quelques ça n'en arrière à la réunion d'abord en Guadeloupe, ensuite nous avons en effet constaté ces problèmes de coefficient géographique et je dois dire que une étude de l'adresse n'est pas inutile, certes, mais enfin quand on sait que les ARS verse une aide exceptionnelle chaque année à la fin de l'année par rapport au fait que le coefficient géographique est insuffisant, on n'a pas besoin d'études, il suffit de faire des comparaisons des budgets chaque année des aides exceptionnelles, chaque année, pour savoir qui allait coefficient géographique, il faut mettre en place, le fait de ne pas donner ce coefficient géographique entraînement immédiatement entraîne en plus une incertitude permanente sur le fonctionnement des hôpitaux dans ces dans ces départements et dans ces territoires, donc je voterai l'amendement. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 1062 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

commission cet amendement vise à permettre aux juridictions financières et aux organismes de contrôle administratif, de contrôler les cliniques privées et leurs sociétés ainsi que des sociétés qui exerce sur elle un contrôle Direct ou indirect en permettant que leur soit transmis les documents comptables et financiers correspondants, il s'inscrit ainsi dans le cadre des mesures de renforcement des outils de contrôle applicable aux structures sanitaires, sociales et médico-social prévu à l'article 32 du présent texte ce contrôle permettra notamment d'identifier les trop-versé par l'assurance maladie, générant ainsi des économies par exemple dans le cadre de l'affaire Orpea : plus de 50 millions d'euros de trop versé avaient été identifiés, je vous remercie. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci madame le président, madame la ministre, chers collègues, de quoi parle-t-on ici, nous avons tous suivi le scandale Orpea au début de l'année, à la suite de la publication du livre les fossoyeurs, ce scandale a conduit à renforcer le contrôle des est pas des des groupes qui les détiennent et c'était une demande de la commission d'enquête de nos collègues Bernard Bonne et Michel Meunier et c'est l'objet de l'article 32 du présent Plfss l'intention de cet amendement à l'intention des des auteurs est clair : faire de même concernant les établissements de santé privés alors plusieurs choses, tout d'abord une observation liminaire, les cliniques privées ne sont pas comparables aux Epad il y avait concernant les pas d'un déficit de contrôles qui tenait notamment différentes sections de fonctionnement fonction soit la fonction dépendance et la fonction hébergement, il y avait aussi un enjeu de tutelle qui sont plurielles et ce n'est pas la même chose concernant les cliniques d'assurance maladie et les agences régionales de santé ont des rôles très claire et identifiés et vouloir contre les établissements de santé oui mais jeter la suspicion non, par ailleurs, si on veut contrôler efficacement les groupes des Epad à moyens constants, on ne peut pas contrôler tout le monde, je crois qu'il faut prioriser il y a une volonté de contrôler les épater et surtout de contrer les les groupes gestionnaires de ces Epad et nous sommes tous d'accord là-dessus, je rappelle également techniques privées sont bien dans le Champ des contrôles au-delà de leur tutelle des juridictions financières, la Cour des comptes peut déjà au terme de l'article L 111 tirer 7 du code des génériques des juridictions financières contrôler les cliniques, elle en a d'ailleurs contrôlée le c'est les chambres régionales et territoriales des comptes le peuvent aussi, en proximité au terme de l'article L 211 va 7 du même code clairement l'amendement ne contrôle pas, il permet de de fournir des des données que la Cour qu'on a déjà quoi, je suis au regret de vous dire chers collègues qui ne fait pas ce que son objet prétend si vous souhaitez que les groupes détenant des cliniques, il faut modifier les 2 articles que je citais à l'instant ici d'amendements, vous portez ne ferait que rendre obligatoire la transmission de documents comptables, or ces informations tout à fait accessible aux juridictions financières qui peuvent exercer leur droit de communication par ailleurs cette transmission des comptes certifiés, a été supprimée pour les établissements contrôlés par la cour à l'occasion de l'ordonnance de mars dernier, la rendre obligatoire pour les cliniques ne semble donc pas cohérent, je propose donc le retrait peut-être de retravailler l'amendement et avoir cette discussion dans le cadre d'un texte sur les établissements de santé, bien évidemment, à défaut l'avis sera défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, la sénatrice le gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement que vous ne déposez madame la rapporteure. Pas de jugement, surtout pas de suspicion, il s'agit bien de proposer que soit permis le contrôle par les juges, direction financière et les organismes de contrôle administratif des établissements de santé privés de leur société satellites ainsi que des sociétés qui exerce sur elle un contrôle Direct ou indirect en permettant que leur soit transmis les documents comptables et financiers correspondants votre amendement transpose et complète pour le Champ sanitaire dans le code de la santé publique, les dispositions qui vont être prises pour les Epad prévu à l'article 32 du PLFSS par conséquent nous amène à un avis favorable à votre amendement. Merci Monsieur, bonne. Oui, madame la présidente, madame Émilie je crois, je crois, effectivement avec Michelle Meunier en a mené l'enquête qui a permis de dire qu'il fallait absolument contrôler les pas des notamment les Ehpad privés habitue créatif tout à fait d'accord parce qu'il y avait effectivement de l'argent public qui pouvait être utilisé de façon anormale par contre, il en est tout à fait différemment au niveau des cliniques et je pense que le gouvernement essaye de rattraper le retard ou l'erreur qu'il a fait en ne contrôlant pas assez ces groupes,

qui ont la possibilité d'être contrôlé au niveau médical, mais qui n'ont pas à être contrôlés sur sur l'arrêt son niveau de l'hébergement hôtelier alors que, au niveau des Epad : ce sont des personnes qui rentre et qui n'ont pas la possibilité de se défendent de la même façon, je crois qu'il fallait effectivement poussé beaucoup plus les contrôles et nouveau des établissements pour les personnes âgées mais ça n'a rien à voir avec les établissements des cliniques, je pense que les contrôles sont exercés aujourd'hui sur le plan médical, ils ne sont pas du tout de la même façon, sur le plan hôtelier, je crois qu'il n'y a pas de raison d'accepter cet amendement telle qu'il est proposé aujourd'hui. Merci Madame Goulet. les fraudes, il est absolument indispensable que l'ensemble des établissements soient soumis au maximum de contrôle parce que l'argent qui est qui est fraudé ne va pas aux urgences ne va pas aux infirmières ne va pas au système de santé, donc moi je vais soutenir très énergiquement cet amendement, pleine d'espoir pour celui que j'ai déposée à l'Arctique. 32 merci madame la présidente, madame le Ministre, moi aussi je vais je vais soutenir cet amendement que j'ai cosigné c'est assez technique des si j'ai bien écouté Madame la rapporteure, malgré tout, vous n'avez pas dit qu'il était satisfait, donc je pense que il y a quand même une possibilité d'aller vers plus de transparence qui qui ne nuit pas, de toute manière, on est dans un contexte un petit peu compliqué pour tout le monde, on s'est rendu compte que des scandales ont éclaté pour les pour les la transparence ne nuira jamais, il n'est pas question d'aller vers la suspicion systématique mais simplement demandé une transparence qui est parfaitement légitime, je vous remercie. Merci madame Meunier. Merci madame la présidente, madame la ministre, j'apprécie l'explication est l'avis favorable que vous donnez à ces amendement comment groupe finir finalement votera d'abord, on était davantage sur une abstention je j'avoue, hein, j'en transparence, mais avec une dissidence donc sur mon collègue co-rapporteur sur le contrôle dans les et Pâques, je pense que c'est de la même démarche et du même principe de transparence qu'il nous faut donc nous nous voterons sur cet amendement, merci madame la rapporteure. Merci madame le président madame le Ministre, mes chers collègues. C'est pas pour ou contre les contrôles. évidemment, sauf que votre amendement telle qu'il est rédigé. Ne fait pas ce qu'il dit c'est tout dans ces cas-là, il fallait modifier les 2 articles que j'ai cité du code de juridique de la juridiction financière, c'est tout, c'est tout ce que je dis. Merci monsieur fier. nous avec notre groupe, on votera quand même aussi cet amendement parce que je crois qu'on a besoin de transparence, on a besoin de redonner beaucoup de confiance entre nos concitoyens et et le système de santé, j'ai bien entendu le l'intervention de notre collègue bonne il y a eu quand même une évolution des cliniques privées, qui au début était l'outil entre les mains des professionnels et qui les rémunérait et maintenant qui passe entre les mains de grands groupes financiers qui cherche aussi à faire des bénéfices et à distribuer des des dividendes et donc ça mérite d'avoir un contrôle qui soit plus appuyé. Merci beaucoup. Je vais, je vais passer au vote. Donc de la maman 697 avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement et je vous demande de bien levé les mains, merci beaucoup, alors qui est pour.

Qui est contre. il est adopté. Alors l'amendement 1140 rectifier du gouvernement.

Madame la présidente, madame la rapporteure donc cet amendement du gouvernement. Propose de décaler à 2024 l'entrée en vigueur des réformes du financement par l'assurance maladie obligatoire des activités de soins de suite et de réadaptation dit SSR et du ticket modérateur, dans le cadre du Ségur de la santé, le gouvernement a engagé une modification en profondeur du mode de financement des établissements de santé, il s'agit de notamment de remplacer progressivement la tarification à l'activité par des modes de financement plus mixte prenant davantage en compte les besoins de santé, la pertinence et la qualité des prises en charge néanmoins sur le Champ du SSR, les établissements de santé et les agences régionales de santé ont besoin de disposer du temps nécessaire à l'appropriation et à la mise en oeuvre des nouvelles modalités de financement pour ce secteur, cette mise en oeuvre nécessite en effet un travail de fond important de la part des acteurs du terrain des ARS et des établissements de santé, ce travail il est, il leur est difficile de le finaliser d'ici la fin de l'année dans le contexte actuel, gestion de crise sanitaire mise en oeuvre de la réforme de la psychiatrie, malgré les importants travaux de préparation et de concertation qui ont été conduits, il convient de s'adapter aux impératifs du terrain, un tel report est donc justifié par la nécessité d'appropriation des nouvelles maligne modalités de financement, j'affirme que notre volonté reste de faire aboutir ses réformes, l'objectif est de redonner des marges de manoeuvre au secteur SSR en terme d'évolution des modalités de prise en charge et de développement d'activités, nous poursuivrons donc bien sûr, les travaux pour assurer la mise en oeuvre pleine et entière de ce nouveau modèle de financement en 2024, c'est pourquoi nous proposons avec cet amendement de décaler l'application du nouveau modèle de financement des soins de suite et de la réforme du ticket modérateur au 1er janvier 2024 je le redis, ce n'est en rien un renoncement ou une remise en cause des objectifs et principes qui ont guidé l'élaboration de ces 2 réformes. il y a pas d'avis de la commission, madame le président parce que voilà l'amendement nous a été communiquée hier soir tard et donc la commission n'a pas pu se prononcer sur cet amendement, donc je m'exprimerai à titre personnel, bon madame la ministre. Cet amendement a le même objet qu'un amendement PLFSS 2022, quand je dis le même objet. Je parle du fond, mais aussi de l'exposé des motifs quasi au mot cet amendement au PLFSS qui reportait 2022 qui reporté d'un an l'entrée en vigueur de la réforme du financement nécessaire avait été déposé le 8 novembre 2021 cette année, nouveau report d'un an avec un amendement proposé le 9 novembre 2022, et que nous discutons ce matin jeudi 10 novembre je ne vais pas une nouvelle fois, revenir sur les problèmes de méthode, Madame la Ministre, mais quand même connaissez nous demander moins de 8 semaines avant la date d'entrée en vigueur théorique, un nouveau report et ce, 2 années de suite aux jours près peut légitimement nous interpelle comment, après plusieurs années de préparation, le gouvernement se trouvait-il encore dans l'incertitude en octobre au point de ne pas inscrire cela dans le texte initial ou à l'Assemblée nationale, nous regrettons l'absence de mesures relatives au financement de l'hôpital dans le texte, et bien nous voilà servis, je rappelle mes chers collègues, que l'on parle de la réforme du financement de SSR depuis le début des années 2007 amendement modifie la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, qui a instauré la T2A, cette réforme a été actée en loi de financement pour 2016 il y a donc sept ans elle devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 après 5 ans permettant sa préparation, je ne sais pas où sont les blocages à quel moment les problèmes techniques évoqués seront-t-il enfin résolu, donc je ne vais pas tourner autour du pot doit tendre à droite, on attend le 8 novembre 2023 report à 2025, comptez-vous un jour mener à bien cette réforme du financement et c'est bien là la question à force de reports, on peut commencer à douter de la volonté du gouvernement d'aboutir, la stabilité n'est pas bonne et elle n'est bonne pour personne. Une observation, vous avez reporté l'an dernier la réforme en supprimant l'année de neutralisation des effets précédent les 3 années de transition, il aurait mieux valu maintenir cette année de neutralisation qui aurait eu lieu en 2022 pour une transition dès 2023, pourquoi ne pas plutôt qu'un report entier rétablir cette année neutralisation en 2023, je constate, je constate que si les établissements privés, pour le coup, en Côte corps très inquiets des effets revenus sur leurs établissements appelé de leurs voeux, ce report, ce n'est pas le cas des établissements publics, les hôpitaux souhaitait bien lancé cette réforme au 1er janvier qui est à travailler, Madame la Ministre, sur des dispositifs transitoires de sécurisation des ressources, vous n'avez pas retenu cette option qui aurait pu être une voie médiane, voilà donc à titre personnel, j'y suis défavorable. Merci, alors donc je vais mettre Monsieur tout de même. Un amendement qui est signifiant, madame la présidente dans quelques mots rapides, moi je, je souscris à que quasiment à l'intégralité du discours de notre rapporteur, mais sauf à la conclusion, parce que cette réforme, effectivement, si on l'applique, comme ça au 1er janvier ça va poser beaucoup de problèmes et donc la sagesse veut qu'on reporte alors après tout, le tous les arguments de Corinne Imbert moi je, hein, et voilà l'historique non, le sujet n'a pas émergé il y a 15 jours, et caetera et caetera, mais la réforme, elle est complexe, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne, voilà et en général, on peut se dire qu'une réforme qui autant reporté, il vaut mieux des fois arrêter les frais et remettre tout à plat, voilà, mais donc ne l'appliquons pas au 1er janvier donc bah faut voter l'avant non du gouvernement. Oui, moi aussi, enfin moi je souscris à la totalité Didier de de l'intervention de la rapporteure Corinne Imbert qu'on parle d'impératifs de terrain quand même, seul un acteur, seule une fédération, à savoir la fédération hospitalière privée demandent ce report et pourquoi le demande-t-elle tout simplement parce que, effectivement, la réforme porte sur la réduction de la part du financement à l'activité, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour un financement plus mixte quand même depuis des années, qui est demandé, en tenant compte des besoins de santé, c'est quand même le point de départ de la pertinence et de la qualité des prises en charge qu'est-ce qui s'est passé, notamment pour la psychiatrie effectivement avant la réforme avec le tarif, la T2A, d'un côté les forfaits global de l'autre, 80 pour 100 des lits ouverts étaient dans les, les, les cliniques psychiatriques privées quoi qu'on pense, parce que moi j'étais un peu dubitatif au départ sur la totalité de de la réforme effectivement donner des années supplémentaires, c'est maintenir cette distorsion un petit peu, je dirais de concurrence du ah, d'un côté une enveloppe fermée et de l'autre des des d'été 2 ans c'est pour ça que de toute façon un façon un an ne suffira pas à la fédération hospitalière privée pour être d'accord avec la réforme, effectivement, c'est une demande forte et quand vous dites de me donner du temps aux acteurs, c'est à cet acteur-là que vous dites, et dans un an, ils ne seront pas plus convaincu, donc effectivement on s'achemine vers un un report si le seul interlocuteur que vous écoutez sur

Beaucoup d'années au moins depuis 2004 que la SSR et psychiatrie demande une réforme du financement de de leurs établissements le les la psychiatrie SSR étant toujours en budget global

pratiquement hier pour aujourd'hui, ce qui empêche évidemment la commission des fins sociales de réfléchir sur le sujet et de se prononcer sur ce sujet, ce qui fait que Madame madame reporter exprimé à titre personnel, je reviens sur le vote de mon abstention, madame, madame la présidente, parce que je crois qu'il est important je j'entends bien ce que demande le gouvernement, par rapport aux cliniques privées, j'entends bien ce qu'a dit Madame la rapporteure sur le fait que c'est peut-être pas l'endroit où il faut le faire, mais ce que ce que je regrette, moi, c'est que hier, alors qu'un amendement avait été proposée pour mieux contrôler de la part de collègues communistes pour mieux contrôler le système de santé privés qui est en train de se mettre en place sur le territoire national d'ailleurs d'être rapportée également par notre collègue médecin de de la région lyonnaise, je crois qu'il faut que nous soyons très. Inquiet et très observateur dans la façon dont actuellement des grands groupes à capitaux privés, et un particulier a avec des systèmes de retraite privées sont en train de prendre la main sur la santé en France, c'est extrêmement dangereux pour la sécurité sociale pour l'établissement public et même pour les libéraux, et donc il est nécessaire, je, je n'ai pas voté parce que je pense que le le la la rapporteure a raison mais je j'ai voté hier l'amendement qui était présenté par nos collègues communistes alertons alertons et et examinons de près ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement dangereux. Merci madame Guigou. Oui merci madame la présidente, je ne voudrais pas cet amendement, voilà, je trouve que c'est regrettable cette réforme est reportée, chaque année, c'est comme la 5ème, branche qu'on reporte et qu'on reporte moi je trouve que, après l'espoir, le désespoir, ça commence à bien faire, donc je ne voterai pas cet amendement.

vers laquelle vis-à-vis de laquelle nous devons être très, très attentif, hein, et notre collègue a fait une remarque c'est plus exactement, les cliniques privées d'hier, cette évolution de regroupement, et donc nous devons être très attentif, mais j'ai une question à poser à Madame la Ministre est-ce que cet amendement résulte d'une difficulté de mise en oeuvre est-ce que c'est un doute sur la volonté politique et puis est-ce que cela se fera un jour, je vous remercie. Merci madame Pumerole. Merci madame la présidente, moi je voudrais insister comme mon collègue Milan sur la marchandisation et la dérive marchande de de notre système de santé qui se fait jour de de plus de façon de plus en plus importante, alors on connaissait effectivement la marginalisation dans le domaine des cliniques privées, je vois sur sur ma région toulousaine quasiment toutes les cliniques privées ont été rachetés à part de qui résistent, j'allais dire par Ramsay Santé et aujourd'hui, le problème c'est grammes c'est monter se s'attaque aussi aux soins primaires et le j'allais dire l'aubaine déserts médicaux et pour eux, une situation intéressante puisqu'il se propose d'installer des cabinets où ils auront des médecins salariés qui sont payés, j'allais dire en fonction du nombre de consultations petits-enfants mieux et plus vite et mieux c'est donc je crois qu'il faut que, vraiment, si on veut préserver notre modèle de santé, il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à cette marchandisation et j'avais posé la question au mois de février à Olivier Véran, qui était alors le ministre a senti, il m'avait dit : on ne peut pas empêcher, empêcher, c'était au moment du de la possibilité de rachat des soins primaires, détenu par la Croix-Rouge, il m'avait dit : on ne peut pas rage empêcher des transactions entre dans le privé, je crois qu'il faut qu'il y a une volonté politique forte au niveau de l'État pour que la marche marchandisation qui est en cours et on le voit tous les jours depuis vraiment envahir tout notre système de santé, je crois qu'on avait un beau système de, de, de protection, il faut le conserver. Merci madame la ministre. je crois qu'on a ouvert de champs Monsieur Mignon a rouvert la discussion mais je crois que l'objet de l'amendement qui a été déposée, enfin qui a été votée, c'est bien celui-là, c'est attention et merci d'apporter, j'allais dire à travers votre abstention une vigilance collective sur les les les risques que vous avez évoquées pour revenir à l'amendement déposé par le gouvernement, moi je vais être très formel, nous n'entendons pas madame la sénatrice. Qu'un qu'une fédération, nous entendons tous les acteurs, et nous travaillons avec tous les acteurs, l'ancienne parlementaire que je suis regrette l'arrivée de certains moments tardif mais pourquoi il arrive tardivement, c'est bien parce que nous essayons et nous avons encore essayer tardivement de travailler pour mettre en oeuvre cette réforme au 1er janvier 2023, force est de constater, et les remontées que nous, qui nous des ARS nous montre le le réel danger de vouloir à marche forcée la mettre en application dès le 1er jeu de janvier 2023 le risque, le risque c'est que, il y aurait une idée, une inégalité d'accès et donc d'effectivité de cette réforme, ce que nous ne souhaitons pas nous souhaitons et je le redis, formellement, je l'ai redit avec force tout à l'heure, mais je le redis avec force, nous souhaitons aboutir sur cette réforme du SSR, elle est, elle elle est légitime, elle est nécessaire, donc nous le faisons, mais nous le nous souhaitons le faire, j'allais dire de façon égale sur tout le territoire et les les signaux qui nous remonte des territoires nous manque de tous les acteurs ne sont pas prêts et donc le risque ne pas voter cet amendement, c'est que cette réforme va se mettre en place, elle va se mettre en place de façon désordonnée, c'est que nous, c'est ce que nous ne souhaitons surtout pas pour une réforme aussi importante et aussi attendu de tous les acteurs et je leur ai je le répète, cette réforme elle est nécessaire, nous en sommes vraiment convaincus. alors je vais mettre aux voix, donc l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Oui : avis défavorable oui oui c'est ça, personnel de la rapporteure, puisque nous n'avons pas pu la l'examiner en commission donc je mets aux voix qui est pour. Qui est contre.

Merci madame la présidente, alors c'est un amendement qui vise à poser le débat au fond de la méthode de construction des lois de finances de la Sécurité sociale, puisqu'il propose de substituer à la logique de la politique de l'offre années des ratios d'analyse financière, une logique de besoins en santé, moi j'étais très content d'entendre 2 fois hier le ministre de la santé, la prévention porter cette idée en en ces termes exacts, nous devons passer d'une logique d'offre à une logique de besoins en santé, je regrette que, alors ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, on va se parler franchement, mais je regrette que, dans ce PLFSS il n'y a aucun marqueur écrit de cette volonté exprimée oralement, encore une fois, par le ministre de la santé et l'objet de cet amendement, c'est bien de d'entamer ce processus de conversion, moi j'appelle le gouvernement à envisager de façon sérieuse qu'en amont du PLFSS de la délibération qu'on a. 2 ou 3 mois avant, en juin ou en juillet, le Parlement soit saisi. D'un document. Pourtant, les objectifs nationaux de santé du pays que le Parlement puisse débattre de ses objectifs nationaux de santé et que, à la suite de ce débat et de l'adoption de ce document, il est l'élaboration du budget du PLFSS voilà, c'est-à-dire que si on ne procède pas si on ne pose pas une méthode d'élaboration différente, on continuera à dire oralement qu'on veut partir des besoins de santé et à nous présenter un texte qui ne porte que une logique d'analyse financière, c'est l'objet de cet amendement. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. Président Madame la Ministre, mes chers collègues, la vocation du plan de 13 milliards d'euros et de soutenir l'investissement et rétablir les capacités d'autofinancement, l'un des critères et donc, notamment celui des ratios d'analyse financière afin de cibler aussi les hôpitaux particulièrement endetté que ces contrats soient assis sur les besoins de santé du territoire est une évidence, l'objet du contrat d'ailleurs précisé à la première phase de l'article 5 ans de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 s'agit au terme de cet article de couvrir la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, si l'intention de Bergeron Jomier d'insister sur la prise en compte des besoins de santé est louable, la rédaction actuelle me semble la satisfaire ne paraît donc pas opportun d'allonger la rédaction de l'article 5 ans de la loi de financement la circuité sociale pour 2021 et donc c'est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le sénateur vous souhaitez dans le cadre de l'article 50 de la Plfss pour 2021, supprimer la référence au ratio d'analyse financière et aux marges financières financières nécessaires à l'investissement et la remplacer par une référence à un nombre de lits hospitaliers, de personnel et de moyens nécessaires à la prise en charge de patients en cohérence avec les besoins de santé de la population, l'objectif de ces mesures, hé bien de redonner aux établissements de santé, les moyens d'investir, y compris en matière d'investissements courants afin d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et de travail des personnels Espitallier je vous rappelle la nouvelle stratégie d'investissement santé est désormais basé sur le projet médical et soignant la validation de ces derniers étant un préalable et indispensable à tout projet d'investissement immobilier, un décret du 30 juin 2021 d'ailleurs précisé les paramètres servant à déterminer le montant des dotations, des besoins de financement nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des soins en priorité par le renouvellement des investissements courants, les besoins de financement nécessaires pour les opérations d'investissement structurant concourant à la transformation du service public hospitalier et enfin les besoins de financement permettant de restaurer les capacités de financement des investissements nécessaires pour garantir la continuité des soins, il ne s'agit donc pas d'imposer des ratios aux établissements de santé, qui en bénéficieront, mais de prévoir les projets les plus adaptées aux besoins de santé des territoires tout en veillant à la soutenabilité financière de ces projets accompagnés par l'État pour ces raisons-là le Gouvernement émet un avis défavorable à votre proposition d'amendement. Merci merci, madame la présidente, madame la madame la Ministre, voilà, j'en profite pour rebondir sur le sujet de des besoins en santé des territoires et de la cartographie parce que je trouve qu'il nous manque quand même un outil d'ailleurs, il y a beaucoup de mesures où on dit on essaye de faire une différenciation entre les territoires sous-dotés les territoires moins sous-dotées, mais il manque quand même un outil précis et moi j'avais déposé un amendement d'ailleurs sur une recommandation de l'Académie nationale de médecine qui disait que il était recommandé d'établir une cartographie sur les besoins en santé des territoires, alors moi j'ai pris un article quarante avec cet amendement, ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que quand on demande un rapport ça passe quand on demande une carte, ça passe pas alors que j'imagine que l'ARS et les ordres en tous les chiffres qui permettrait d'établir une cartographie et donc je la demande et je de je j'informe que je reçois chaque année un Atlas démographique de la profession vétérinaire qui est très utile, alors je ne vois pas enfin, ou alors ça existe quelque part, mais il faudrait qu'on puisse me le fournir merci. C'est madame la rapporteure générale. merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, moi je comprends comment les inquiétudes de de mon collègue Jomier, cependant, je ne vais pas soutenir son amendement, mais je voudrais dire que on a jamais tant dépensé en France pour la santé et pour autant on se trouve face à lits qui ferme ah mécontentement sur tous les territoires, enfin je je passe les détails, et je pense qu'il faut effectivement y travailler en amont, j'ai eu l'occasion, quelques jours avant l'examen de de ce PLFSS d'en parler aussi avec les les collaborateurs de de Bercy, hier nous avons vu avec le ministre, il y a une intention de travailler un peu plus tôt et et je crois qu'il faut que nous aussi on se voit dans la proposition et que, avec les ministres, on essaie de de réfléchir bien avant, parce que c'est un sujet très honnêtement qui dépasse les clivages politiques, on a tous des réponses à apporter à nos territoires à nos concitoyens et et je crois vraiment fermement que, il faut s'y prendre vraiment beaucoup plus tôt pour essayer de faire en sorte que toute cette masse budgétaire objectif national de dépenses de l'assurance maladie, hé bien puisse l'expliquer bien le dépenser et en tout cas qu'il réponde aux problématiques que l'on n'a, sur le terrain et qu'on entend partout. Oui merci madame la présidente, c'est un amendement qui est extrêmement intéressant et qui rejoint d'ailleurs tout ce qui a pu être dit et par les uns et par les autres en discussion générale je je voudrais juste ajouter elle je ne voterai pas pour des raisons que que vous pourrez comprendre c'est que en fait il nous faut maintenant réaliser que si nous continuons dans le même système, l'ensemble du système de santé va dans le droit dans le mur, il nous faut donc réfléchir, comme le disait Bernard Jomier et au financement et à l'organisation territoriale de de notre système de santé et à beaucoup d'autres choses, par ailleurs, l'organisation d'hôpital et cetera, et cetera parce que nous avons tous dit, alors il est important Madame la Ministre, de ne pas perdre de temps supplémentaire, donc il est important que dans les semaines à venir, je ne dis même pas les mois à venir, mais que dans les semaines à venir, des réflexions soient mises en place entre le Parlement et le gouvernement les les différents syndicats et associations concernées afin que nous puissions travailler et sur le financement de la Sécurité sociale et sur l'organisation territoriale de la santé et sur l'organisation des hôpitaux et sur l'organisation de la médecine d'aval des hôpitaux, et caetera et caetera, il y a beaucoup de choses à faire, à remettre en place et je crois qu'il est nécessaire que nous fassions cela non pas d'une façon globale, en plus, sauf dans la réflexion mais loi par loi de manière à ce que nous ne soyons pas ensuite noyé dans des amendements type alcool ou type de tabac qui empêche de de réfléchir complètement sur différents sujets. Merci Monsieur Chassaing. Oui, madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, moi je suis plutôt favorable à cet amendement parce que on se rend compte que, dans certains territoires, on est obligé de garder des des services à notamment les services d'urgence et d'autres services indispensables si vous voulez au territoire alors qu'il y a pas énormément de population mais on est très éloigné de CHU ou même de d'un CHR où on est un petit peu rattaché à à un CHR qui, notamment au niveau obstétrique fait enrôler pour la néo-natalité c'est dans ce d'hôpital qui est quand même très excentré, faut le conserver, mais il faut l'interpréter, si vous voulez ces besoins là c'est pas en fonction de la population, ni peut-être aussi de la fréquentation, c'est en fonction du territoire pour que tu te demander la même accès aux soins, donc l'ARS effectivement déjà le fait mais c'est pas mal de de le de le noter. Merci Monsieur Jomier. Je vais décevoir Daniel Chassain, parce que j'ai retiré l'amendement en fait parce que, évidemment, vous l'avez compris, c'était un amendement qui visait à ouvrir le débat et qui visait à ce que j'ai dit au gouvernement et pour faire suite à à l'intervention d'Élisabeth Doineau je mettons cette proposition sur la table, faisons précéder la séquence budgétaire du PLFSS qui a lieu à l'Automne par une séquence, juin, juillet, je ne sais pas que 2 ou 3 mois avant, qui permettent de débattre sur des objectifs nationaux de santé publique et de les adopter et nous mettrons comme ça les choses en ordre, nous discuterons d'abord de nos priorités de santé le processus d'élaboration ne devrait partir des territoires remonter nationalement être validé au Parlement et ensuite le gouvernement construit la ligne budgétaire, c'est la bonne façon de redonner sens à nos politiques et de redonner de la compréhension à ses lois de finance de la Sécurité sociale qui sied noms apparaissent de plus en plus comme étant la simple duplication d'analyse financière et votre réponse était parfaite, Madame la Ministre, sur ce que le le descriptif de ce qui se passe actuellement, mais ça n'est pas la bonne méthode pour notre pays. Merci donc l'amendement est retiré l'amendement 65, même de la commission, même la rapporteure. Merci madame le président madame le Ministre, mes chers collègues, cette. Combien par le présenta le présent amendement d'apporter une sécurité juridique à la garantie de financement qui prendra fin au 31 décembre 2022, il s'agit également d'interpeller le gouvernement sur l'opportunité de dispositif transitoire à l'issue de cette garantie, alors que le niveau d'activité notamment en médecine chirurgie obstétrique demeure en 2022 encore inférieur à celui de 1019 les ressources des établissements demeurent fragilisé ou voici l'objet de cet amendement. Madame la présidente, madame la rapporteur tout d'abord répondre à Monsieur Millon et Monsieur Jomier Monsieur Millon sur les enjeux de gouvernance et de financement. Je vous invite à participer au CNR en santé, qui sont organisées, dont ces 2 thèmes sont des thèmes majeurs et sur lequel à la fois les parlementaires à la fois les associations d'élus, à la fois les, les, les établissements participent donc je vous invite à y participer, comme à aller dans les territoires, en ce qui concerne l'organisation territoriale et et la réponse à apporter aux besoins de santé des c'est des CNR territoriaux, je peux vous assurer que c'est assez passionnant de travailler à la fois avec les élus, les personnels soignants et nos citoyens qui participent à ces CNR il en ressort des idées très intéressantes, mais sur les enjeux de l'hôpital sur les enjeux de gouvernance et de financement, il y a un CNR national qui est organisé sur ce thème et donc vous serez effectivement et si vous le souhaitez, le bienvenu pour y participer, madame la rapporteure le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement. Qui propose d'inscrire dans la loi la prolongation au second semestre 2022, la garantie de financement pour les santé donc face à la crise sanitaire et c'est qu'on se fait conséquences financières, le gouvernement a immédiatement apporter une réponse dédiée et adapté au travers de de textes au second semestre 2022, le dispositif de garantie de financement a été prolongé par un arrêté ministériel visant à la mise en oeuvre opérationnelle des mesures de la mission flash pour les soins urgents et non programmés pour l'été 2022 au titre des mesures d'urgence, d'organisation et de fonctionnement du système de santé cet arrêté avait lui-même comme base légale : l'article L. 31 31 du code de la santé publique, pour ces raisons je suis défavorable à votre proposition d'amendement Merci madame la présidente, hé bien nous le groupe écologiste soutiendra cette l'amendement de de la rapporteure parce que, effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les hôpitaux publics, par exemple, la fait FHF la la signaler ont pris 80 de nouveau d'ailleurs des hospitalisations de la Covid 80 % alors que je le rappelle, ils n'ont que 60 % en termes de parts fin d'activité, donc 60 % de MS, et donc, effectivement, ils sont encore à 5 % de moins, enfin ils sont encore en sous, sous-activité de 5 % par rapport à l'année 2019 qui était l'année de référence avant-Covid là je j'ai pas revenir sur tout à l'heure, mais effectivement, la fédération hospitalière privée, elle qui n'a pas eu autant de, enfin de déprogrammation, bien entendu, puisque elle a, elle, a pris qu'une partie de des hospitalisations Covid a dépassé déjà effectivement l'activité de 2000 19 et donc ne souhaite pas une mesure transitoire de lissage en quelque sorte, reporté encore sur 2023, mais moi je pense qu'il faut effectivement eu égard quand même au service public Keran pour la prise en charge de la Covid, les établissements publics, hé bien effectivement avoir encore une période transitoire pour pour ceux-ci, au moins jusqu'en 2023. Merci madame la rapporteure.

Donc, que dit l'amendement d'abord, il vient faire 2 choses : d'une part sécuriser juridiquement ce que vous faites, par simple arrêté, c'est quand même pas rien, donc pourquoi cet avis défavorable, je peux vous donner la l'arrêter si vous le souhaitez, de loi d'urgence ou permettait déroger jusqu'en juillet dernier, aux règles de financement et de mettre en oeuvre cette garantie de financement, ce n'est plus le cas depuis le 30 juin que vous le vouliez ou non, or il s'agit de la troisième année de dérogation au droit commun, ce n'est juridiquement pas souhaitable cet avis défavorable, donc incompréhensible, vous vous opposez à vos propres mesures, si c'est cela, j'attendais un tout petit peu mieux de la vivant la bienveillance du gouvernement, d'autre part, cet amendement avait un objectif d'appel les établissements n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité 2000 19 et n'est pas certain qu'en 2023, il le retrouve, nous ne sommes pas favorables à une garantie de financement ad vitam eternam, évidemment il ne s'agit pas de revenir à la dotation globale mais quid, donc des ressources pour 2023, les hôpitaux ont besoin de visibilité pour leur gestion et nous attendons. Cette visibilité avec eux, voilà pourquoi je continue à maintenir cet amendement bien évidemment. Merci, alors je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est donc adopté l'amendement 734 monsieur Iacovelli. Oui, madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le code de la sécurité sociale ta différents différentes catégories d'établissements de santé en fonction desquels il aurait attribué une échelle tarifaire correspondant à l'ancienne dotation globale dite ex ou une échelle tarifaire ex-au les catégories d'établissements visés par les dispositions B et C de cet article permettent l'attribution d'une telle d'une échelle tarifaire, ex-DG sont historiquement fermé cependant comme tous les établissements publics de santé, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les explique participent au service public hospitalier à ce titre, il est demandé au gouvernement de remettre au Parlement un rapport portant sur la possibilité des explique ex-Hawk uen de basculer à l'échelle tarifaire, ex-DG et l'impact d'une telle bascule. Merci madame la rapporteure votre avenir. Si Madame le président, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc c'est une demande de rapport, donc c'est ça l'avis défavorable de la commission non, moi je suis intéressée par les explications de la Mini sur l'éventuelle possibilité pour certains établissements de basculer dans un autre, riz, je vous remercie. Merci madame la Ministre, l'avis du gouvernement. la possibilité pour ces établissements relevant de l'échelle tarifaire dicte ex-oh que viennent d'effectuer un changement pour l'échelle d'ex- DG, il s'agit déjà d'une échelle tarifaire commune pour l'ensemble des établissements qui était auparavant sous-dotation globale qu'ils soient publics ou privés à but non lucratif, tout compris intègre la rémunération des personnels médicaux, salariés de ces établissements, à la différence des établissements fonctionnant avec des praticiens libéraux qui facturent directement leurs honoraires, il est donc légitime de pouvoir différencier les tarifs hospitaliers en fonction des conditions d'exercice des personnels médicaux et par conséquent en fonction des catégories d'établissements pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement, à défaut, j'y serai défavorable. Non non il il n'est pas retiré, je le maintiens, par principe, notamment parce que nous avons un amendement qui a été rejetée article 45 sur la question des explique et je pense que c'est un vrai sujet, la question des explique aujourd'hui dans notre pays représente 8 pardonnez-moi de, d'avoir une explication de vote, madame la présidente, mais les explique représente 8 % de l'offre de soins dans notre pays et c'est le parent pauvre aujourd'hui et on le voit dans un certain nombre de territoires et notamment dans le mien à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, nous avons un vrai problème d'égalité de de remboursement des soins pour les explique et donc, je maintiens mon amendement. Qui est contre pas adopté après l'article 25 toujours, mais un pont c'est moche pour le 800 66. Demain. Oui merci madame la présidente, alors c'est un amendement d'appel puisque c'est un rapport de demander au gouvernement d'étudier le lancement d'un plan d'urgence pour la psychiatrie, l'absence de la psychiatrie dans le PLFSS est préoccupante en regard de la situation de ce secteur, j'avais pointé dans la discussion générale de la psychiatrie de la pédiatrie, bon ben la pédiatrie à ces mesures. Ponctuel d'urgence, on attend peut-être quelque chose sur la psychiatrie de même ordre, mais ça ne sera pas suffisant car depuis les années 1980 malgré une augmentation de la population générale, les moyens pour la psychiatrie ont non seulement peu évoluer mais ont souffert de la fermeture de 2 tiers des lits d'hospitalisation, la psychiatrie, parent pauvre de la médecine est aujourd'hui un secteur sinistré qui nécessite une refondation que les assises organisées par le gouvernement, ce printemps, non pas destiné pour une meilleure prise en en soins des patients, il s'agit d'améliorer les conditions de travail des soignants de lutter contres les mesures privatives de liberté, faute de moyens humains suffisants et de garantir le respect, donc des droits fondamentaux des individus et des patients, le secteur psychiatrique doit être conforté comme l'échelle de proximité de prise en soins et également comme modèle d'organisation pour la santé, l'investissement public dans la psychiatrie dont la pédopsychiatrie, proche de l'effondrement, on revient un petit peu aux aux enfants, doit permettre l'ouverture de lits nouveaux et de structures où et surtout de structure ouverte pour prendre en charge les patients et permettent le recrutement et la formation du personnel qualifié, l'urgence est donc de rebâtir un secteur psychiatrique public apte à prendre soin tous les patients sur l'ensemble du territoire, et ce, en respectant, je l'ai dit tout à l'heure, les droits fondamentaux et la dignité des personnes soignées, cet amendement demande un rapport évaluant les coûts et les bénéfices enfin d'un véritable plan ambitieux pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatre. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. Demande de rapport Madame le président, c'est un avis défavorable. La ministre de l'avis du gouvernement. Donc des demandes un rapport un avis défavorable, néanmoins je comprends bien l'intérêt des questions donc, pour les 6 amendements concernant les 6 rapports un avis défavorable et je m'engage à vous apporter une réponse écrite à la question qui est la vôtre. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 866 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour, qui est contre qui s'abstient, adopté le 1064 madame Laoui Merci madame la présidente, madame la Ministre, c'est un amendement d'appel de notre groupe, socialiste, écologiste et républicain, qui a été travaillé avec la CFDT EFS mais qui est largement partagée partagée et qui vise à la remise d'un rapport au Parlement sur l'état de l'établissement français du sang, les personnels de l'établissement français du sang, nous lance un cri d'alarme et ce cri d'alarme à de grandes conséquences sur la baisse des ressources de sang et de plasma d'ailleurs il y a également un appel d'urgence vitale à la mobilisation pour augmenter ses ressources, mais en fait il y a un véritable problème d'un d'attractivité, le personnel de l'EFS donc lance un préavis de grève du 22 septembre au 2 janvier afin de dénoncer la situation catastrophique de l'EFS et demander des moyens nécessaires pour assurer la mission essentielle qui leur est confiée, l'EFS n'arrivent pas à recruter n'arrive pas à fidéliser les personnels après 13 ans de non-révision des classifications et bientôt quatre position sur 10 en dessous du SMIC, ceux qui y travaillent le font dans des conditions très difficiles, je ne parle pas des heures supplémentaires qui sont accumulées par les personnels, notamment ceux qui sont affectés à l'activité d'immuno-hématologiques délivrance 51 pour 100 des salariés du prélèvement dépasse les 12 heures d'amplitude de travail c'est 42 % de l'activité immuno- immuno- hématologiques délivrance donc ce que nous proposons c'est une revalorisation salariale de l'ensemble des professionnels, alors que la prime Ségur a été refusé à ces derniers une révision de la classification des rémunérations à hauteur des enjeux de la mission du service public des effectifs suffisants, une amélioration des conditions de travail, si nous voulons préserver ce modèle éthique français de transfusion si nous voulons préserver ce service majeur pour le bon fonctionnement de nos hôpitaux et une bonne prise en charge des patients, nous devons et vous devez agir vite. Merci, même la rapportant je vous demande d'être vraiment concis. néanmoins, pour votre information Madame le Ministre, sachez qu'il y a eu beaucoup d'amendements proposant de relever la dotation pour l'établissement français du sang, ces amendements ont été déclarées irrecevables de l'article 40 pour autant la question de l'équilibre financier de l'établissement français du sang et des moyens pour assurer sa mission que nous savons, indispensable, est au coeur, est au coeur du sujet, donc peut-être que vous nous apporterez à d'autres occasions, des éclairages et tout ce que souhaite faire le gouvernement sur ce sujet-là promesses. Merci madame la ministre. Madame Lauvergeon comme je me suis engagé je vous apportera une réponse écrite à la question que vous posez, néanmoins le le le l'enjeu de l'Établissement français du sang a aussi été discutée les collègues députés ont aussi beaucoup abondé dans ce sens est un enjeu majeur sur lequel nous avons déjà apporté des moyens supplémentaires sur lequel nous bien sûr 25 millions d'euros à alors, poursuit le le l'engagement, le financement de l'établissement de l'EFS à hauteur de 25 millions de donc c'est un bel engagement mais néanmoins, nous savons qu'il y a aussi des problématiques structurelles sur lequel nous allons travailler avec l'EFS et un problème en plus des problèmes éthiques structurelles, nous savons aussi qu'il y a des problématiques de personnel soignant et de nombres de personnel soignant, donc c'est un enjeu majeur et nous partageons tous le même objet. Madame brûlant. Merci madame la présidente, madame la Ministre je nous faisons partie de ce qu'a évoqué Madame la rapporteure, c'est-à-dire d'amendement de notre groupe, qui ont été retoquée au titre de l'article 40 tout à fait dans l'esprit que vous avez évoquées mais nous soutiendrons l'amendement de notre collègue parce qu'effectivement j'entends ce que vous venez de dire à Madame la Ministre, sur votre prise en compte de l'établissement français du sang, mais on est quand même dans une situation extrêmement inquiétante parce qu'on, je ne reviens pas sur les conditions de travail qui ont été très bien développé à l'instant, mais on en arrive à une situation où on est obligé d'annuler des collectes de sang alors que, par 2 fois ont été lancés, des appels d'urgence aux dons du sang puisque nos stocks, on le sait bien, ne sont pas au plus haut, donc je voudrais insister à mon tour sur la nécessité de revalorisation salariale, il y a des salariés qui sont encore aujourd'hui en dessous du SMIC et donc si on veut rendre attractifs ces professions, il y a évidemment et puis derrière, tout ça sans dramatiser, parce que je crois que chacun y est attaché, mais il y a notre modèle français du don du sang, avec toute sa vocation éthique et le refus de la marchandisation de ces médicaments ou de ces dispositifs dérivés du sang et je crois que cet effort doit conduire au maintien de ce modèle auquel nous tenons tout ce temps. Merci madame Ferré. Merci madame la présidente, madame la Ministre je soutiendrai bien évidemment cet amendement, je souhaitais aussi apporter ma contribution, mais les arguments pour expliquer ce ce choix, je voudrais tout d'abord relayé les propos de la directrice générale de l'ESF qui dit nous voulons mieux prendre en charge les patients défendre notre modèle éthique améliorer notre souveraineté sanitaire il nous faut des moyens en investissements importants et un fort soutien de l'État, alors les personnels sont mobilisés, ils alertent sur le besoin de postes supplémentaires, cela a été dit, les conséquences sont nombreuses sur la collecte et après la crise sanitaire et bien on voit que ce nombre est encore trop faible, l'ESF est confronté ainsi une double pénurie à la fois médicale et de dons et c'est aussi la Fédération française pour le don de sang bénévole qui alerte dans son au cours de son dernier congrès, elle alerte sur la situation de l'le et la nécessité de le doter en moyens humains et financiers pour faire face aux besoins qui sont indispensables et je voulais relayer auprès de vous, ses soutiens et ses demandes. Merci même président, alors ça a été en partie dis moi je voulais relever comme il y a actuellement je crois 300 postes vacants dans cet établissement. Comment effectivement le paradoxe où on annule des collectes de sang et en même temps à la radio, on entend des campagnes urgentes d'appels d'appel donc là on est vraiment faute des d'années durant, de non-revalorisation, on est dans un cercle vicieux postes vacants et

donc mail intérim et comme on va barrer l'intérim maintenant la conséquence, ça va être la fermeture de services voire d'hôpitaux de maternités, faute de personnel parce que on sera allé au bout du paradoxe et du cercle vicieux de la crise d'attractivité, donc il faut mettre fin quand même à des années de déflation salariale et en plus, dans pour le l'établissement là d'avoir été en quelque sorte les oubliées du Ségur fait vraiment que c'est la goutte de de trop dans la crise d'attractivité. Merci madame la présidente, madame la Ministre, c'est l'occasion également de se pencher sur la situation dans les outre-mer, j'ai eu plusieurs fois évoqué les plus problématiques liées à la transfusion sanguine sur mon territoire, mais aussi lors des auditions du président de l'EFS au niveau national, j'ai eu l'occasion d'attirer son attention sur certaines de ces problématiques et il est également question aujourd'hui de la situation de la Guyane en Guyane, il y a pas de collecte, les raisons pour lesquelles les collectes avait été supprimé en Guyane non non plus aucun objet dans la mesure où le diagnostic biologique pour les concernant les difficultés qu'il y avait à l'époque ne sont plus un sujet donc il faudrait également prendre en compte cette situation parce que les dons du sang en Guyane sont ou bien parce qu'il y a en ce moment avec la Guadeloupe le EFS, Guadeloupe, Guyane et des dons qui viennent de la Guadeloupe, mais beaucoup aussi viennent de d'ici de de l'Hexagone et la difficulté, c'est que c'est le développement des maladies auto-immunes, que ça va générer à long terme pour certaines personnes, notamment pour les personnes drépanocytaire pour lesquels il faut de faire des dons réguliers, donc c'est un sujet, je vous demande aussi de faire en sorte que les collègues reprennent en Guyane c'est important. je voudrais juste vous informer, j'ai encore cinq demandes de prise de parole, alors si vous pouviez être concis, Madame la Ministre, il faut surtout entendre que on a besoin d'une loi santé parce que les collègues tous les collègues ont vraiment raison sur beaucoup de points, je crois que c'est vraiment un appel au secours, merci merci, madame la présidente, en fait, on ne devrait pas discuter de l'EFS en Plfss puisque théoriquement c'est un financement d'État sauf que, il y a une dotation de l'assurance maladie, ce qui fait que on peut raccrocher la discussion. Qui est décroissante, c'est une dotation qui date de il y a quelques années et le le chiffre que vous avez donnée madame la mini-je je ne sais pas lequel c'est si c'est celui de la dotation de la licence maladie mais je crois que il va passer à 10 millions d'euros et théoriquement c'est un financement qui doit s'éteindre, résultat, la direction de l'EFS est obligé de serrer les boulons et donc effectivement il ne peut pas y avoir de progression salariale pour les agents et donc il y a un découplage avec d'autres agences sur des postes similaires en termes professionnel et deuxièmement, il y a une restriction des frais de collecte, c'est le premier problème, le second c'est que l'EFS vend au LFB. Et ils vont aux hôpitaux, enfin, ça passe par le LFB mais il ne peut pas vendre au prix qu'il souhaite et donc il est obligé de vendre à des prix qui ne couvrent pas suffisamment ses coûts, bon maintenant, il est urgent d'apporter des réponses, parce que le système notre système français est en train de souffrir durement, ça a été dit par mes collègues et donc je vais, je vais être bref, donc nous allons maintenir bien sûr cet amendement et nous allons demander que chacun se prononce dessus vous, on ne peut plus et ce qui fait le sujet, et parfois il y a des demandes de rapport qui valent plus que des amendements portant directement modification d'un article du PLFSS. Merci, je vous signale qu'il aura un scrutin public sur sur cet amendement et même la rapporteure générale. Oui, il faut pas s'étonner, on se mobilise tous, pour l'établissement français du sang, parce que le sang c'est la vie et que on ne peut pas intervenir dans beaucoup de situations, si on n'a pas cette ce ce ce volume de sang à proximité je pensais intervenir à l'article 45 parce que, tout comme Bernard Jomier vient de le dire, je pensais qu'effectivement une partie des financements arrivent par le le le Fonds de modernisation et d'investissement, santé et donc c'était à ce moment-là que je voulais intervenir et non pas sur ses cet article comme vous le faites je je soutiendrai pas forcément votre article, mais tout ça pour dire que, en réalité, c'est très important qu'on suive vraiment comme le lait sur le feu, les, comment les volumes de sang et qu'on puisse financer cet établissement, moi j'étais intervenu à un moment où le Ségur a fait encore un oublié c'était justement cet établissement parce que bah pour recruter du il faut qu'on puisse les rémunéré au même niveau qu'on les rémunère ailleurs alors c'était pas le cas pour l'établissement français du sang, je pense qu'il faut être très très attentif parce que c'est vraiment le le coeur de la vie quoi et je, je, je pense que nos collègues ont raison en tout cas de de Maistre le débat sur cet établissement parce qu'en tout cas nous on y est très sensible, merci.

à ce que vous répondiez de manière laconique en nous disant que vous allez nous répondre par écrit, c'est pas une succession de questions écrites, c'est un débat et, dans le cadre de ce débat, j'ai une question à vous poser, il y a 40 % du personnel de cet établissement public qui touchent moins que le SMIC, c'est tout à fait. Inadmissible, c'est pas possible que dans un établissement public aussi crucial que celui-là, une telle proportion de personnel touche moins que le SMIC à quelle échéance pensez-vous atteindre ce niveau du SMIC qui est un niveau minimal pour l'ensemble des personnels et quel crédit comptez-vous affecté dans les délais les plus rapprochées pour que les personnels touchent au moins le SMIC.

il y a personne ici qui peut penser qu'on va résoudre le problème par un rapport, hein, et donc c'est pas parce que on va voter contre cet amendement que on est pas préoccupé par la santé de l'EFS d'autant plus, je le répète que c'est un symbole,

Oui, madame la présidente à la ministre, il ne vous aura pas échappé que je ne serais pas d'accord avec mon collègue Olivier Henno, qui viennent s'exprimer parce que, puisqu'on ne peut pas demander quoi que ce soit pour l'EFS au travers notamment de la sanction de l'article 40 nous nous rabattant vers un rapport alors je sais bien qu'un rapport, ça ne règle pas tous tous les problèmes, mes chers collègues, mais ça permet au moins de savoir ce que le gouvernement a l'intention de faire par rapport à toutes les critiques que vous avez évoqué les uns les autres donc soyez cohérents, vous ne pouvez pas, à un moment dire ça marche pas pour le FN, ça, ça se ça craque de partout, les personnels n'en peuvent plus et nous n'assurons pas la mission de service public qui est potentiellement donc supporté par cette structure et et ne pas savoir exactement ce qu'il se passe, donc nous en cohérence et au travers donc de cet amendement, nous proposons et au travers des scrutin public, vous allez pouvoir vous prolongez nous proposons un rapport, je sais bien qu'il y a une jurisprudence sur les rapports, comme l'a rappelé hier, notre collègue sur sur l'article 40 quarante-cinq mais à force de refuser toute forme de débat, hé bien, c'est le parlementarisme qui est mis en question question aujourd'hui, y compris dans cette haute assemblée. Mais si, alors donc j'ai été saisi, comme je vous l'ai dit, d'une même un ministre oui. Je crois que nous partageons tous ici. La volonté de garder le système éthique d'abord du don du sang et donc il dit : la volonté de garder le système éthique de don du sang, madame la sénatrice, hein, dit accompagner l'EFS l'EFS est actuellement comme. Tous les professionnels de santé, vous l'avez signalé madame la sénatrice se dire soumis à des problématiques d'attractivité des métiers, des personnels soignants et pour aller moi très souvent comme chacun d'entre vous dans un établissement, nous savons bien que là nous avons un réel problème de recrutement un réel problème de recrutement qui est. Qui êtes aussi du. Alors je m'étonne des chiffres que vous donnez, je ne crois pas qu'en France on puisse être payé en dessous du SMIC dans les proportions donc on va regarder ce problème, et en tout au en tout état de cause, une mission IGAS IGF a été lancée sur le financement de l'Établissement français du sang, parce que je le redis, la volonté du gouvernement, hé bien de conserver ce modèle éthique du don du sang qui ici je crois nous et tous si cher. Merci, alors donc je vais lancer le scrutin public qui a été demandée, donc par le groupe socialiste, donc sur l'amendement numéro 1064 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement va être cédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Le résultat du scrutin numéro 45 soixante-quatre compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 330 pour l'adoption 107 contre 223 le Sénat n'a pas adopté et je passe à l'amendement 1104 Merci madame la présidente, madame la Ministre, ne me dites pas qu'il s'agit d'un rapport c'est nous connaissons tout à fait les raisons et les réponses simplement cet amendement, nous l'avons travaillé avec les fédérations et les associations représentatives des personnels qui oeuvrent dans le domaine de l'action sociale et je vais appeler cet amendement si vous le permettez, amendement des oubliées du Ségur en effet les établissements et services sociaux médico-sociaux et de santé associatifs font face, vous le savez très bien à une insuffisance de professionnels du fait des difficultés pour recruter et conserver les salariés dans ce contexte, le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire a octroyé à juste titre des revalorisations salariales dans certains secteurs, mais malheureusement pas dans d'autres, créant ainsi des différences entre par exemple le secteur public et le secteur privé à but non lucratif et donc associatif, je crois que chacune et chacun d'entre nous, a été interpellé dans nos différents départements par cette question des disparités encore entre les champs de la santé, les personnels des des personnes âgées et des personnes handicapées et le secteur de l'action sociale ou encore les soignants et les autres professionnels l'indispensable, je pense par exemple aux chauffeurs qui transportent les usagers dans les établissements, et caetera au sein d'une même association et je pense que nous avons été nombreux à être interpellé sur ce point dans la même association certains salariés sont les Z'oubliées du Ségur, d'autres ne le sont pas, donc ce n'est pas justiciables, ce n'est pas justifiable, eu égard à l'engagement de l'ensemble de ces professionnels, donc nous demandons bien sûr un rapport mais Madame la Ministre, nous sérieux encore plus heureux d'obtenir de votre part une réponse et des échéances. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. Demande de rapport, donc c'est un avis défavorable de la commission madame. Madame la ministre, avis du gouvernement. Madame la présidente, madame la rapporteure, vous proposez que soit remis au Parlement arabe. Pour évaluer la réalité d'augmentation des rémunérations des métiers du soin du médico-social et du social, permise par le Ségur de la santé ces revalorisations décidées dans le cadre du Ségur de la Santé et des suites représente un effort historique qui représente 11 milliards dans l'Ondam, en 2023 et bénéficier un nombre très important des professionnels du secteur sanitaire et médico-social, le gouvernement assume également d'avoir parfois cibler ces mesures sur les métiers dont le manque d'attractivité, était le plus criant, les sujets relatifs aux évolutions du secteur, notamment en lien avec l'attractivité des métiers ont fait l'objet de nombreux travaux ces dernières années, permettant l'élaboration de stratégies concertées d'acc très activités notamment dans le secteur du grand âge et de l'autonomie, ces travaux ont vocation à être approfondie dans le cadre du programme prioritaire du gouvernement relatifs au recrutement et à la fidélisation des métiers des secteurs sanitaires et sociales, au regard de l'ensemble ces ces éléments, je suis défavorable à votre amendement. Merci Monsieur Chassaing. Oui, madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, bon alors effectivement, comme l'a dit Monsieur sur je ne sais pas si l'amendement ne va pas régler les problèmes, mais il faut quand même dire que ça a été d'ailleurs très bien exprimé dans une association, un n'est pas d'un donc tout le monde va être pris en charge pour les 183 euros plus même davantage pourrait être soignante, je voudrais dire que ce qu'a fait le gouvernement revalorisation moi je trouve que c'est, c'est très bien et je me félicite pour ça, si vous avez dans la même association, une maison d'accueil spécialisée et que vous ayez des gens qui ont participé aux soins mais qui font fonction d'aide-soignante, ils ne sont pas pris en charge le le secrétariat non plus les personnes qui s'occupe donc de l'environnement ou des bâtiments non plus, alors qu'en Ephad, c'est le cas à côté, vous avez un foyer occupationnel qui est pris en charge par le département, effectivement, c'est le département qui en a la charge et il faut bien sûr que l'État Vienne en aide aux départements : je crois que c'est prévu mais tout ça, si vous voulez, il faut quand même que ce soit clarifiée parce que on a des personnes qui travaillent dans la même association mais dans dans un établissement différent qui veulent changer pour aller dans un autre et dans un autre établissement, donc il faut effectivement coordonner tout ça merci. Merci madame Meunier. Merci madame la présidente, l'amendement que vient de présenter notre collègue Jean-Pierre Sueur et juste, je ne voterai bien sûr et je rajoute le secteur des médecins territoriaux dans le secteur de la protection maternelle et infantile et de la santé sexuelle, le précédent gouvernement, Madame la ministre avait affirmé en avril dernier, y compris pour ses médecins concernés dont je viens de parler que ces primes avait, je cite, vocation à être transformé lors des prochaines lois financières, nous y sommes en complément de traitement indiciaire afin de pouvoir, pouvoir être prises en compte dans le calcul de la retraite cet été le PLFR ah bien converti la prime Ségur en complément de traitement indiciaire pour l'ensemble des personnels soignants de PMI à l'exclusion des médecins, on parle là de 1700 médecins de PMI et des médecins de santé sexuelle, l'attractivité de la médecine de PMI en dépend, on la connaît, elle est bien inférieure à celle d'autres cadre d'exercice de la médecine salariée je rappelle que le traitement en début de carrière et les 2500 euros les rapports paieront le rapport de la Cour des comptes ont souligné le préjudice de la désertification médicale des PMI pour les bébés, les femmes, les jeunes et les familles, le ministre a insisté sur son attachement à la prévention médicale hier lors de l'article 17 qui a été débattu ici le 1er rendez-vous de prévention intervient lors de la visite prénatale assuré par les PMI, faisons donc en sorte que ces médecins territoriaux soient pleinement pleinement soutenus dans leur mission par rapport au rapport, je crois que si nous faisons le total des demandes de rapport qui n'est pas encore fait, dans le cadre de ce Plfss mais uniquement sur la branche retraite il y a demandes de rapport, donc si on prend les branches, une par une, on arrivera facilement à une centaine de demandes de rapport, nous savons très bien que cette demande de seront jamais exaucé, nous savons très bien que plus on demande des rapports au Gouvernement moi on en aura, on en demande déjà pas beaucoup et on n'en a que d'une culture que 30 % à peu près qui sont réalisés, alors c'est le sujet qui a été abordé par monsieur Sueur est un sujet extrêmement important, mais nous pourrions directement le prendre à notre compte,

depuis le début de l'année 2022 les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux font face à une inflation sans précédent depuis des décennies qui pèse fortement sur leur situation financière, cette inflation estimée à environ 6 dans les dernières prévisions de l'Insee pour 2022 masse d'importantes disparités d'évolution des prix, notamment ceux relatifs à l'énergie pour lesquels une hausse est envisagée autour de 30 ce sont des perspectives inquiétantes, loin de l'évolution initialement prévu la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2022 intégré une hausse des prix aux environs de 1 un véhicule 5 % pour 2000 vendus la hausse réelle pourrait être 3 à 4 fois supérieure à 7 perf cette perspective donc il s'agit Madame de voir. Pour ces établissements une augmentation pour l'année à venir et dans le cas du effet Merci l'avis de la commission madame la rapporteure défavorable, défavorable, madame le président, merci madame la ministre. Donc l'amendement 872 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour qui est contre qui s'abstient donc pas adopter un moment 690 même Procaccia. Oui, il s'agit aussi d'une demande de rapport mais qui attire l'attention sur les Français qui n'ont pas de médecin traitant et donc qui demande un rapport sur les pénalités financières qu'endurent ces assurés sociaux.

En fait c'est un amendement qui concerne la prise en charge de la fibro magie au titre de l'affection de de longue durée, c'est une maladie qui est très invalidante et donc ce que je propose, c'est que dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation, il puisse y avoir. Un rapport sur cette sur cette merci, madame la rapporteure, l'avis de la commission des favorables, madame le président si Madame la Ministre, même avis je mets aux voix donc l'amendement 695 défavorable de la commission et du gouvernement qui. Pour qui est contrat qui s'abstient pas adopté à l'article 25 bis, la maman 66 madame la rapporteure. Merci madame le président, madame la Ministre, chers collègues, c'est un amendement de suppression parce que cet article concerne les règles d'autorisation d'activités de soins d'équipements matériels lourds qui ne relèvent pas d'une loi de financement de la Sécurité sociale. Merci la vie de du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, madame rapporteure votre amendement propose du supprimer l'article 25 beef relatif à la simplification de la mise en oeuvre de la réforme des autorisations d'activités des soins et d'équipements matériels lourds qui ne relèvent pas d'une loi de financement de la Sécurité sociale, le 1er volet de cet article permet au groupement de coopération, de porter une autorisation d'activités de soins sans être érigés en établissements de santé, pour mémoire, l'une des orientations de la réforme des autorisations, a été de transformer certaines autorisations d'équipements de matériels lourds en autorisations d'activités de soins cette disposition vise à ne pas déstabiliser les coopérations mixte public-privé existantes et évitera ainsi la multiplication des titulaires d'autorisations d'activités de soins pour contenir le nombre de ml et les dépenses d'assurer associé le second volet de cet article rétabli la durée de vie initiale de 7 ans les autorisations d'activités de soins dont les conditions d'implantation et techniques de fonctionnement ne seront pas réviser, il permet également aux ARS de déroger temporairement à l'obligation de solliciter l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins pour certaines demandes d'autorisation sur la base de critères d'offre de qualité et de sécurité, sécurité des soins qui seront définies par décret en l'absence de mesures, le traitement de l'ensemble des autorisations concernés ne pourra être pris en charge à moyens constants, par les établissements de santé et les ARS elle induirait également un décalage de la mise en oeuvre de la réforme des autorisations d'au minimum un an, décalant d'autant l'impact financier associé cette mesure, en plus d'écarter les risques qu'un retard pris dans le renouvellement et l'octroi de nouvelles autorisations ferait peser sur l'offre de soins et la sécurité juridique des établissements de santé présentent un réel impact sur les dépenses d'assurance maladie, justifiant sa place en loi de financement de la Sécurité sociale pour l'ensemble de ces raisons je suis défavorable à votre avis. Merci, alors je vais mettre. Aux voix l'amendement 66 de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Bien la qui est contrat

qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'article 25 quater Madame Cohen pour une prise de parole. Merci madame la présidente, là, l'article 25 Water prolonge jusqu'au 31 décembre 2000 le dispositif permettant aux médecins et aux infirmiers de travailler jusqu'à 72 ans, dans les établissements publics de santé l'intention du gouvernement de prolonger cette dérogation face aux besoins du de personnels médicaux et paramédicaux est en quelque sorte une mesure de sauve qui peut entre 2017 et 2019 le d'ombres, de Saint-, âgés entre 70 et 72 ans, a progressé de 15 % par an, la solution ne peut être de prolonger la génération du Baby boom le plus longtemps possible en attendant l'arrivée des nouvelles générations de personnel, nous en avons longuement discuté hier, Madame la Ministre, il faut former plus de médecins et donc donner des moyens aux universités Monsieur Brown, ministre de la Santé et des solidarités, disait hier que les mesures prises par le gouvernement, permettaient de former plus de médecins et il paraissait assez satisfaits de ce résultat, mais moi je veux tempérer son enthousiasme 11000 médecins sont formés chaque année à peu près le même le même nombre qu'en 1975 alors que la population a augmenté de 20 % avec des besoins en santé, qui sont beaucoup plus importants, pourquoi, parce que tout simplement la la population qui vieillit et plus nombreuses voilà et présentent davantage de poly-pathologies permettre aux médecins et aux infirmières de travailler jusqu'à 72 ans, n'est pas sérieux et n'est pas à la hauteur des besoins en terme de santé, c'est ce que je nous voulions dire avec mon groupe, à l'occasion de cet article, je vous remercie.

si par exemple vous êtes dans un service à l'hôpital et tout fonctionne parfaitement, hé bien vous avez 70 arbres est obligé de partir, par contre, vous allez en clinique au fait ma heureusement les beaux jours de la clinique et en même temps vous vous supprimez un praticien qui qui fonctionne parfaitement à l'hôpital, donc je suis, je pense, effectivement, cet amendement n'est pas adapté à ce qui se passe actuellement, et moi je ne voterai pas favorablement à cet amendement il faut au contraire essayer pour les médecins qui sont en bonne forme physique, hé bien, qu'ils puissent continuer leur action jusqu'à 72 ans.

article 25 inquiets ça même Cohen. Oui, madame la présidente, cet article, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale porte sur les praticiens à diplôme hors Union européenne, les pas du alors que la mission flash sur les urgences, pointait la nécessité de prolonger l'autorisation d'exercice, aucun article n'était prévu dans le projet de loi initial sans cet article 25 qui inquiète de nombreux établissements auraient mis un terme au contrat des au 1er janvier 2023, ce n'est pas la première fois que nous évoquons ici la situation des pas du et malgré la loi de 2019, leurs difficultés à exercer demeure je vous ai moi-même adressé un courrier en tout cas pas à vous, Madame la Ministre, bien Monsieur le Ministre, fin septembre pour vous alerter sur les conditions d'accès au statut de praticien praticien associé notamment pour celles et ceux qui doivent passer les épreuves de validation des connaissances, les pas du nom lauréats des EVC de 2021 sont priés de repasser leurs épreuves en 2023, mais sans aucune précision sur le calendrier exact pour les 2 voies d'accès procédure dérogatoire au concours les où concours les ARS et le Centre national de gestion chargé d'examiner les dossiers d'autorisation d'exercice sont très en retard, laissant les professionnels dans une attente et une incertitude ingérable, malgré leurs compétences et leur expérience et médecins sont beaucoup moins rémunérés que leurs collègues assistant et praticien hospitalier ces médecins, sages-femmes, pharmacienne, pharmaciens, chirurgiens-dentistes dont le nombre est estimé à 4000 sont devenus au fil des ans des éléments indispensables pour le fonctionnement des hôpitaux, y compris hospit'au hospitalo-universitaire aussi aberrant que cela puisse la grande majorité de ces palu sont aujourd'hui en situation irrégulière en matière de droits de au séjour à l'heure où la tension est maximale dans les hôpitaux, dans les EPHAD cette situation est inacceptable et, d'ailleurs le ras le report proposé à avril 2023 par notre collègue Jomier et pour lequel un avis favorable de la commission a été donnée est certes une respiration mais il faut aller beaucoup plus loin, nous allons soutenir aussi notre collègue

non membre de l'Union européenne ayant travaillé en France se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire mais cette attestation d'pour qui permette le recrutement du praticien, le temps que l'examen de ce de son dossier par la commission d'autorisation d'exercice détermine s'il pouvait s'inscrire à l'ordre mais c'est déterminer s'il avait besoin de formation complémentaire ou s'il devait cesser sa pratique bien elle était valable jusqu'au 31 décembre 2020 la déjà été prorogée en dix jusqu'au 31 décembre 22 en septembre 22, la majorité des praticiens, la vient d'être dit, étaient toujours en attente de l'examen de leur dossier par la Commission nationale, plus de 4000 dossiers ont été déposés et l'organisation retenue, à savoir un entretien Oral de chaque candidat par la commission d'autorisation d'exercice ne permettra pas l'ensemble des praticiens inscrits dans cette procédure de régulariser leur dossier et de le voir afin de sécuriser l'exercice de ces professionnels et l'organisation des établissements, cet amendement vise donc il a décalé au 31 décembre 2023 la date de validité des autorisations temporaires, alors pourquoi pas seulement un an, mais pourquoi décembre 2023, je dirais, par précaution, nous proposons un délai jusqu'en décembre pour nous laisser la possibilité que j'espère nous ne t'utiliseront pas d'y revenir dans le prochain PLFSS s'il y a encore lors de de du prochain des commissions qui ne l'ont pas été matériellement tenue.

disons-le, un problème de procédure, elle est beaucoup trop complexe et la preuve en est que se multiplient les cas personnel qui nous sont remontés ou quand on les regarde, on dit non c'est pas normal et puis la procédure est très stressantes d'ailleurs pour les concernés, qui je le rappelle, sont des professionnels de santé qui exercent dans notre pays, parfois depuis longtemps, donc moi je vous invite au delà de cet amendement de report de quelques mois pour examiner les dossiers qui s'empilent actuellement à nous proposer, Madame la Ministre, une procédure plus simple et soyez sûrs qu'on l'examinera avec beaucoup de bienveillance. Merci, alors l'avis de la commission, même la rapporteure. Si le président le ministre un avis défavorable sur le 954 et un avis favorable sur 1094. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure, permettez-moi de vous faire une petite explication avant de donner un avis défavorable sur les deux amendements parce que nous devons. Traiter les pas du et nous parlons bien des pas du gestion stock j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ici lors d'une réponse de questions au gouvernement, je n'aime pas ce terme, mais c'est le terme qui était dans la loi, c'est-à-dire nous parlons bien là des professionnels qui sont, qui exerce avant la loi votée en 2019 nous avons depuis le mois de juillet, traiter un très grand nombre des dossiers qui étaient en stock, il était aux alentours de 4000 il nous en reste, nous en avons traité près des 3 quarts il nous reste à peu près le quart restant, nous proposons de pouvoir traiter ces dossiers avant le 30 avril et nous avons les moyens et nous avons mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le faire, ça ça concerne la première partie, sur lequel il faut aller vite apporter une réponse à ces praticiens dont nous avons besoin et d'assurer, pour eux, la lisibilité de l'exercice de leur exercice professionnel, ça c'est la première partie, et elle est importante et je le redis, nous avons été en mesure grâce à l'Ordre des médecins, grâce aux ARS et grâce au Centre national de gestion de mettre les moyens pour traiter un grand volume de dossiers qui n'a pas, n'avait pas pu l'être en 2020 à cause de la crise sanitaire puisque les membres du jury sont des professionnels de santé,

ce pourquoi nous vous proposons le 30 avril c'est bien pour régler cette première partie de la loi, c'est-à-dire la gestion des professionnels dit de stock, maintenant, vous avez raison de souligner qu'il y a une 2ème, procédure qui a été votée dans le cadre de la loi, ce sont des professionnels qui sont rentrés après la loi, et donc là on on traite des professionnels dits de flux sur ces flux, une première partie de ce qu'on appelle les EVC, a été faite en février 2022, nous sommes en train d'analyser les conséquences de cette façon, façon, faites par la loi, d'évaluer les nouveaux, les nouveaux pas du et nous sommes en train de réfléchir à des modalités d'assouplissement, notamment dans le cadre du délai du stage de 2 ans et nous reviendrons très vite vers vous pour assouplir la gestion de ce flux pour ne pas recréer un stock du flux mais aussi pour des problèmes à ces praticiens d'avoir une visibilité sur leur avenir et à voir pour les hôpitaux une lisibilité aussi sur le l'employabilité de leurs professionnel, donc je ne suis vraiment pas favorable à l'allongement du délai, je pense qu'il faut rester, il faut se fixer des objectifs et je prends l'engagement qu'ils seront tenus, nous avons été capables en 6 mois, de traiter une grande majorité il faut vraiment régler au plus vite cette partie du stock, vraiment, je le redis pour pouvoir très vite se mettre et ce que ce que nous faisons de façon simultanée en ordre de bataille pour gérer le flux et surtout à porter des modifications dans le cadre dans un cadre législatif pour améliorer la prise en charge du flux et puis nous sommes aussi soumis de demande de créer de création de de pas du pour d'autres professions, vous l'avez évoqué et nous serons peut-être en mesure de travailler aussi dans ce domaine, donc vraiment un avis défavorable je crois que ce serait un très mauvais signal envoyé en allongeant le délai, j'assume parfaitement la responsabilité de dire qu'au 30 avril nous serons en mesure d'avoir réglé cette première partie, qu'il faut régler le plus vite possible. Merci Monsieur. Juste en un mot, Madame la Ministre, nous on souhaite aussi qu'au 30 avril toute avril tout soit réglé, donc il y a aucun problème, par contre, je ne te souhaite pas avoir au mois de mai, des gens qui viennent nous voir en nous disant : ah bah oui, mais pour telle raison, hein, et puis maintenant, ministère, on nous dit la date est dépassée, donc c'est tout, voilà nous on, on, on souhaite cette souplesse de quelques mois supplémentaires mais ont souscrit à votre objectif, bien sûr, et cela même mon Oui merci madame le président ben je tiens compte de ce que vient de de dire madame la ministre, et par contre je retire mon amendement, mais au profit de celui de Bernard Jomier. Merci monsieur lévrier. Oui merci madame la présidente, juste un mot très rapide tout à l'heure on parlait de délai qu'on voulait reporter pour la loi, et cetera, là, le gouvernement s'engage à respecter une date, envoyant un signal clair et ne changeront pas, ne donnons pas encore un signal contraire contraire pour dire on peut donner encore un petit peu de temps au cas où, non, il y a des engagements, il faut les tenir et c'est très important de les tenir. La présidente. Et juste attirer votre attention, madame la ministre sur une visite que l'on a fait l'hôpital de cette année, l'hôpital de Lafontaine il y a un vrai problème avec les sages-femmes à diplôme étranger qu'il faut absolument traiter c'est autre chose, ça ne ne sont pas les pas du j'en suis bien consciente mais néanmoins je voulais attirer votre attention sur ce sujet. Merci, alors je vais mettre l'amendement 1094 qui a reçu un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté je mets aux voix, l'article 25 inquiet, ce qui est pour contrat qui s'abstient, il est donc adopté même la présidente. Bon, les débats sont très intéressants et loi de moins de l'idée tous les les restera notamment, il nous reste 270 amendements, je vous rappelle que nous finissons à 18 heures ce soir que nous reprendrons vendredi matin non, samedi matin, j'espère que nous serons aussi nombreux, samedi matin, mais ce que je demande quand même, c'est si on ne veut pas ouvrir le samedi soir, le samedi, la nuit et on ne veut pas ouvrir le dimanche, d'essayer d'être un peu plus concis dans la présentation des amendements, je veux dire les, les, les objets, on les a sous les yeux, relire ligne aligne tous les objets de toutes les lignes de l'objet, je veux dire on peut faire une synthèse, je veux dire on est habitué à faire des synthèses, je pense qu'on on a la capacité de le faire et d'être un peu plus concis dans les prises de parole, je sais que ce n'est pas, c'est pas bien de dire ça et que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse mais néanmoins je pense que si on pouvait terminer samedi dans l'après-midi, je pense que ça arrangerait tout le monde, on a une semaine pour le PLFSS un vrai sujet, quand on a une quand on a 3 semaines sur le PLF pour un budget qui est quand même un peu différent et ce serait bien, terme peut-être qu'on ne colle pas des âgé au moment du PLFSS. Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, monsieur le président du Sénat a reçu de madame la première ministre transmission du projet de loi de finances rectificative pour 2022 dès ce mercredi 9 novembre dès lors et après concertation avec les groupes politiques et la commission des finances, nous pourrions avancer le délai limite de dépôt des amendements de séance initialement prévu le mercredi 16 novembre à 12 heures au mardi 15 novembre à 17 heures il y a-t-il des observations, il en est donc ainsi décidé, je vais suspendre la séance et la séance sera reprise à 14 heures 35 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.